L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finance adoptée par l'Assemblée nationale pour 2021. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 43.

l'article 43 prévoit que les recettes de la part ex taxe des espaces naturels sensibles de la taxe d'aménagement puissent être affectés à la renaturation des friches urbaines et sols pollués. C'est naturellement une tâche absolument nécessaire et le génie écologique est évidemment une piste très intéressante pour un tendre l'objectif du zéro artificialisation nette mais la renaturation des friches et lors des pollutions particulièrement coûteuses et risque d'absorber une part majoritaire de ces retraits or cette part de la taxe d'aménagement constitue aujourd'hui la principale recette affectée à la biodiversité et aux espaces protégés leur financement public risque donc de baisser les départements n'ont pas été consultés sur le sujet et sont particulièrement inquiets de cet article 43, comme l'a rappelé l'AFD, ils estiment eux aussi que, alors que les dépenses croissantes du RSA pourrait déjà rogné les Budgets alloués aux espaces naturels sensibles gérés par les départements fléché cette taxe dédiée à la biodiversité, vers de la dépollution urbaine très coûteuses pourrait inspirer une grande partie des ressources dévolues à la biodiversité est ce que cela est opportun, le président de la République a annoncé à plusieurs reprises, une augmentation des surfaces protégées en France la stratégie européenne de la biodiversité de l'Union européenne et la stratégie nationale des aires protégées prévoit la même chose la France s'apprête à accueillir à Marseille le congrès mondial de la nature et un G20 sur la biodiversité, va se tenir aussi la COB de la Convention sur la diversité biologique importante puisque devant fixer les objectifs à 2030 et puisque la France a annoncé vouloir y jouer un rôle diplomatique, seuls 20 % des files Natura 2000 sont en bon état de conservation d'où le risque de contentieux européen à terme et les moyens affectés à la protection de la biodiversité sont très faibles en France. J'ai assisté à un colloque, il y a quelques mois sur la renaturation c'est fantastique ce que la science de la, de l'écologie peut fermer un coût exorbitant, évidemment, Monsieur le Ministre, on aura besoin d'être rassurés sur le fait que cette taxe, la part de la taxe à l'envers, la biodiversité, sera bientôt, mais dans l'enveloppe ne compte, le compte n'y est pas merci. Un amendement en 77 Monsieur Féraud, bon madame Préville pardon. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme l'a fort bien dit mon collègue Joël Labbé vient, elle vient de le dire, la taxe d'aménagement et la principale recette fiscale affectés à la biodiversité en France, en élargissant les possibilités d'usage des recettes de cette taxe à de nouveaux postes de dépenses aussi justifié soit-il, le risque est grand de voir diminuer les recettes de la taxe affectée aux espaces naturels sensibles et en particulier aux aires protégées, la biodiversité, ce risque est d'autant plus important que les nouveaux postes de dépenses introduit par l'article, à savoir notamment la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbaines sont extrêmement coûteux, certains départements intéressés pourraient ainsi y consacrer une part importante voire majoritaire entraînant une diminution délétère du financement actuellement, dédiés à la protection de la biodiversité, l'anticipation des effets d'une telle disposition, semblant faire largement défaut et les risques étant considérable, il nous apparaît raisonnable de la supprimer le temps que le gouvernement mûri sa réflexion, on en est un, en analysant finement les tenants et les aboutissants de telles dispositions, rappelons qu'à défaut d'obtenir une augmentation une sécurisation des financements actuels pour la protection de la biodiversité, doit être une condition sine qua non pour financer la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbaines, le mécanisme du fonds friche à l'issue du conseil de défense écologique du 27 juillet dernier semble tout indiqué le gouvernement a toute latitude pour augmenter en conséquence l'enveloppe qu'il a initialement souhaité fixer à hauteur de 300 millions d'euros, je vous remercie. Je demande le retrait de cet amendement, madame la sénatrice d'une réforme qui est motivée par 2 éléments, finalement vous dites où je vais dire la même chose que vous vous dites la même chose que moi, on n'arrive pas tout à fait à la même conclusion d'abord, vous savez que cette cette part départementale de la taxe d'aménagement, fait l'objet d'une sous-consommation chronique dans un grand nombre de départements et d'ailleurs plutôt dans des départements à dominante urbaine, donc le fait de d'offrir la faculté, vous l'avez dit, la possibilité de de travailler à des opérations de renaturation de terrain laissés en friche, me paraît s'inscrire pleinement dans les objectifs que vous avez appelé de vos voeux, deuxièmement. les moyens dédiés à la lutte contre l'artificialisation des sols, l'ampleur des opérations de construction et d'aménagement finalement lié et responsable de cette artificialisation je pense que ça mérite à travers cette réforme cette, je leur ai dit cette faculté qui est donc,

il est plutôt un appel pour dire les départements avec cette taxe d'aménagement ont globalement consommer davantage et appelle peut-être à augmenter cette part, voilà l'objectif qui est poursuivi, raison pour laquelle je demande le retrait. C'est le président, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur a été précis dans ses propos et je les partage, il a rappelé ce qui animait la présentation de cet article dans le projet de loi de finance tels que nous vous le présentons et il a aussi rappelé que cela relevait de la possibilité et non de l'obligation, il a enfin souligné que les niveaux de consommation de certains se relatifs à certains sous objectifs rendait tout à fait tenable cette mesure sans contrarier les objectifs notamment rappelé par le sénateur abbé donc l'avis est défavorable à cet amendement. amendement. Il est maintenu, donc vais mettre aux voix, cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adapté. Un amendement en 27 présenté par monsieur le rapporteur. Je mettre aux voix, quels sont ceux qui sont pour, qui sont contre, ils s'abstiennent adopté je suis saisi de deux amendements identiques. Qui font l'objet d'une discussion commune le 100 93 ans, et le 927 pour le 193 Madame loisirs. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc cet amendement permet aux organes délibérants des communes ou des EPCI d'exonérer de la taxe d'aménagement en tout ou partie les parkings qui font qu'ils choisissent l'option du revêtement de sol drainant cette technique conjugue remplissage gazon est remplissage pavés afin de répondre non seulement aux usages mais aussi d'introduire davantage de végétalisation dans les espaces urbains, ce type de Parking à plusieurs fonctions environnementales infiltration verticale des eaux restauration des échanges des échanges air-terre au lustre contre les îlots chaleur. Aménagement de cheminements piétons pour des parkings vers comme par exemple les grandes surfaces commerciales et végétalisation en milieu urbain au regard donc des enjeux et des nombreuses externalités positives qui bénéficie à l'ensemble de la collectivité, il est à mon sens important de soutenir cette technique par une fiscalité adaptée et dans les meilleurs délais pour répondre et notamment aux enjeux climatiques et écologiques. Oui, je défends le l'amendement de notre collègue Daniel Gremillet, comme l'a dit non. Collègue hein, cet amendement vise à octroyer la possibilité aux collectivités territoriales et leurs groupements d'exonérer de la taxe d'aménagement en tout est parti, les constructions Aménagement de surfaces de stationnement perméable, un revêtement drainant qui permet de lutter contre l'artificialisation des sols, ce faisant, il s'agit de soutenir les collectivités dans leur effort de végétalisation au regard de nombreux bénéfices qui résulte de cette politique publique, lutte contre les îlots de chaleur urbains, la pollution et les inondations, préservation de la biodiversité de la qualité de l'air, contribution à la santé physique et mentale et au bien-être des personnes, amélioration du cadre de vie. Alors, la vie c'est une demande de retrait et je vais m'en expliquer. Il s'agit, en fait, le par l'article 43 et par votre amendement. Vous. Finalement, vous allez à l'envers de la réforme que défend l'article 43, il s'agit en effet de créer une incitation fiscale à la création de places de stationnement qui sont situés, ça c'est l'article. Au-dessus ou en-dessus dessous, pardon, des immeubles afin d'éviter, dans un 1er temps le déploiement parfois, je le dis quelque peu intempestifs. Des parkings en extérieur et où, à côté des habitations, alors bien sûr, et je partage pleinement ce que vous avez évoqué les les arguments pour dire effectivement un Parking végétalisé ombragés avec même des parfois des, des, des fossés drainant des seuls drainant c'est bien largement souhaitables à l'imperméabilisation encore trop souvent rencontré notamment dans lesquels on ne laisse que une ou 2 espèce d'arbre qui végète parce que ils sont complètement enserrée dans l'imperméabilisation mais je rappelle que cette d'abord ça vise aussi à, de, de, de mandats d'artificialisation et surtout ça permet, ça doit permettre une meilleure utilisation des espaces de Parking pour permettre aussi aux villes, il faut le dire de densifier raisonnablement là où il y a des espaces pour l'habitation, de manière à retrouver plus de d'espaces verts et de nature dans certains endroits, finalement par des poches qui ne soient pas des poches de Parking mais des poches de véritables espaces verts pour travailler à la qualité de vie et je pense pour ma part qu'il faut dans un 1er temps laissé cette réforme se mettre en oeuvre avec une exonération unique, sinon on aura un manque de lisibilité et je vous mets mon billet au feu que il se passera une chose, vous aurez des parkings qui seront en ouvrage mal utilisés et vous aurez d'autres parkings végétalisés de meilleure qualité que certains mais qui seront aussi sous-utilisé et donc on y perdrait en lisibilité en efficacité de la dépense publique. C'est le même avis, monsieur le président, c'est un avis défavorable pour les raisons évoquées par monsieur le rapporteur, je ne les reprend pas je partage aussi l'objectif de stabilité et de laisser un peu de temps à cette réforme et cette fiscalité avant de la modifier, c'est la raison pour laquelle tant sur les propositions qui sont portées dans ces amendements qui, sur les propositions d'exonérer de suppression d'exonérations qui viennent au de modulation de la taxe d'aménagement, l'avis du Gouvernement est défavorable au nom de cet attachement à la stabilité et à laisser vieillir un peu si vous me permettez cette expression la la réforme de la taxe d'aménagement, donc ça sera défavorable pour ces raisons-là sur les autres. Je veux mettre aux voix, ces 2 amendements identiques, quels sont ceux qui sont pour. Que sont ceux qui sont contre.

Quels sont ceux qui sont contre. Il n'est pas adopté.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement propose de supprimer l'abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal pour les entrepôts et en gare non ouverts au public, faisant l'objet d'une exploitation commerciale fait l'article 43 prévoit que les, les recettes de la taxe d'aménagement puissent être affectés à la renaturation des friches urbaines et sur l'pollué c'est fort souhaitable, mais c'est très coûteux et ça risque d'absorber une part importante des de ses recettes, avec un abattement sur la taxe d'aménagement, c'est des financements publics en moins pour mener cette tâche fondamentale, est ce que c'est au portant dans la même période, où le le président de la République, ça a été dit déjà ce matin, a annoncé qu'il fallait augmenter les surfaces protégées en France que le gouvernement s'apprête à publier sa stratégie nationale des aires protégées et qu'aujourd'hui seulement 20 % des sites Natura 2000 Français sont en bon état, donc je vois là une contradiction entre les objectifs fixés par le gouvernement et les moyens mis en place la biodiversité étant sous-financé actuellement et cet abattement risque encore de dégrader cette situation financière merci. Le doux 79 Madame Préville. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais faire un petit rappel au sujet de la biodiversité. C'est que nous connaissons une baisse drastique à la fois en espèces et en c'est à dire en qualité et en quantité absolument vertigineuse et nous n'avons pas vraiment encore commencé à endiguer ce phénomène l'artificialisation des sols et l'une des grandes causes de la disparition de la biodiversité en France 9400 % du territoire était artiste artificialiser en 2015 et la consommation d'espace croît en moyenne de 1,4 % par an depuis 1992 ceci entraîne une perte d'espaces naturels, agricoles et forestiers, mais également une disparition des fonctions biologiques du sol une perte des systèmes des services éco-et un danger finalement pour nous, la France est engagée au travers du plan national biodiversité à lutter contre l'artificialisation des sols, la fiscalité représente un des moyens pour atteindre cet objectif cependant certains outils fiscaux vont à l'encontre de cette ambition et constitue ce qu'on appelle une subvention néfaste pour la biodiversité, que la France est engagée pourtant à réduire progressivement ces aides fiscales sont encore nombreuses et très peu d'actions ont été entreprises pour respecter cet objectif pourtant en 2020 constitue une date butoir pour la France, objectif d'Aïchi congrès mondial de la nature ou la France va devoir faire valoir les mesures qu'elle a adoptée pendant ces dernières années et le projet de loi de finances et le dernier point possible pour avancer sur ces objectifs, ces assistants fiscales ont un double impact, elle représente des dépenses pour l'État et les collectivités, et sont en partie facteur de dégradation de l'environnement et de perte de biodiversité dans le contexte actuel, où les Français ont exprimé au travers du grand débat leur souhait d'entamer une véritable transition écologique de protéger l'environnement, mais également de voir baisser la fiscalité et le niveau d'imposition la subsistance de ces aides fiscales est un non-sens cet abattement ne fait pas sens au vu du rythme d'artifice allusion d'artificialisation des sols pardon croissant, comme je l'ai mentionné ni au vu de la perte monétaire que cela engendre pour les collectivités, départements et régions, cet amendement demande donc la suppression de cet abandon, cet abattement, je vous remercie. monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, cet amendement a été particulièrement bien bien défendus par nos 2 collègues Guillaume Chevrollier et Angèle Préville je rajouterai, monsieur le président, monsieur le ministre, que plus ça va, moins ça va dans la politique du en même temps on on ne peut pas vouloir préserver la la biodiversité et l'environnement et continuer un développement économique à tout crin, en particulier vers les zones d'activités extérieures, comme ça a été dit, les grandes surfaces, le E-commerce, on ne peut pas ce type de mesures incitatives avec absolument contre- contre- productif par rapport aux politiques que l'on doit mener donc je le défends également avec force. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc je vais reparler de l'artificialisation des sols et elle entraîne une perte de, comme je l'ai dit des espaces naturels, agricoles et forestiers, chaque année, le CEREMA étudie son impact indique que la dynamique ne faiblit pas, cet amendement vise en conséquence à supprimer l'abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes lorsque ses locaux ont été construits sur des sols qui n'était pas encore artificialiser dégage s'est engagé, comme j'ai, je l'ai dit tout à l'heure au travers du plan national biodiversité à lutter contre ce phénomène, le gouvernement entend réduire les niches fiscales ayant un impact défavorable sur l'environnement, cet abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et en gare non ouverts au public en fond. Alors une demande sur identique sur tous les bancs, je vais donner la réponse qui est une demande de retrait et je vais là encore donner quelques éléments d'appréciation pour expliquer les raisons pour laquelle je ne suis pas favorable, j'estime en effet que, et vous l'avez évoqué de la même manière modernisés, rénovés étendre des locaux commerciaux, ça ne conduit pas nécessairement à une artificialisation des sols, je m'explique : de plus en plus on voit aujourd'hui dans des zones d'activités ou des zones commerciales des mutations d'espace ou de bâtiments pour reconfigurer et c'est vrai également en ville, ce qu'on appelle la ville qui se reconstruit sur elle-même et parfois même pas toujours, je ne vais pas non plus être naïf en redonnant je dirais des espaces plus aérés, avec davantage de de présence de nature et des débuts, il faut le dire aussi de construction donnant beaucoup plus de place au végétal et au bon fonctionnement naturel et écologique des espaces, raison pour laquelle

pression démographique qui continue d'exister dans un certain nombre de territoires, y compris urbain, je rappelle que l'abattement de 50 % pour les cons ce pour les actifs abritant les activités économiques pour par des constructions, a été mis en oeuvre en 2010 et qu'il avait à l'époque pour objectif de ne pas alourdir la fiscalité des acteurs économiques par rapport au régime de la taxe locale d'équipement je rappelle aussi, et vous le savez que parfois quand vous êtes entre 2 territoires voisins de périmètre d'intercommunalité, ça amène des concurrences stériles et ou inutiles, voilà ce que je ce que je voulais donner comme élément je veux également dire qu'il faut faire attention à certains des effets de bord, donc je le redis, je partage pleinement, et je pense d'ailleurs que si un amendement devait être adopté, ce serait plutôt le 12 37 puisque le 12 37 explique bien que ce sont des espaces actuellement des espaces de nature, on va le dire, donc, dans le cadre de la l'ambition du gouvernement de zéro artificialisation nette il y aurait là une logique. L'avis du gouvernement. Monsieur Chevalier. merci Monsieur le Président, malgré les arguments toujours très pertinent du rapporteur général je vais maintenir mon amendement parce que je, je considère que, aujourd'hui, cet abattement, il profite surtout à à la à la grande distribution ou aux entrepôts surface de logistique et ce sont elles, d'ailleurs qui artificialiser beaucoup et et sont bénéficiaires de cet abonnement et donc là au nom d'une justice fiscale, c'est cet amendement, lui il est là pour rééquilibrer un peu les choses vis-à-vis du petit commerce, c'est la raison pour laquelle je je le maintiens. monsieur l'abbé. puisqu'on veut re centrer les commerces sur les centre-villes ce qui est évidemment d'avenir et ce qui est demandé par nos populations, on ne peut pas en même temps elle favoriser en extérieur en périphérie en périphérie urbaine dans ces endroits que le l'urbaniste David Mangin qualifiait dès 2004 de métastases péri- urbaines, merci. il nous faut avoir le courage ou je ne sais pas comment on peut le qualifier de vraiment changer les choses, il faut faire des efforts et et ça ne se fera pas sans et et sans fin, je ne sais, enfin je sais pas comment exprimer voilà donc on se doit de faire parce que les choses ne changent pas et on est face à une baisse de biodiversité qui n'est pas enrayée, jusqu'à présent donc, vraiment, et c'est une petite mesure celle-ci mais il faut vraiment y aller Donc, je vais mettre aux voix, ces amendements qui ont reçu un avis de retrait de la commission et un avis défavorable du Gouvernement quels sont ceux qui sont. Quels Quels sont ceux qui sont contre. Ils sont adoptés. Ils sont adoptés et le 12 37 tombes. Je suis saisi de deux amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune le 14 10, monsieur l'abbé. Oui, cet amendement a été proposé par France urbaine, le code de l'urbanisme permet aux communes et EPCI de fixer le taux de la taxe d'aménagement entre 1 et 5 % selon les aménagements réalisés dans différents secteurs, il leur permet également de majorer ce taux jusqu'à 20 % dans certaines zones, en cas de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d'équipements publics généraux l'article 43 du présent PLF prévoit notamment d'élargir les motifs d'employes de la taxe d'aménagement majorée et donc les secteurs d'application du taux toutefois afin de ne pas pénaliser, voire de promouvoir l'installation d'activités en centre-ville par exemple, en rez-de-chaussée d'immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allégement de la fiscalité de l'aménagement, le présent amendement vise donc à autoriser les communes ou EPCI qui recourent à la majoration de facultatif de taxe d'aménagement à prévoir une augmentation différente pour les logements et pour les locaux d'entreprise afin que l'impact de la majorité majorations de taux soient adaptés aux caractéristiques de chaque marché, il s'agit ainsi de permettre le financement des équipements publics, sans mettre en cause l'équilibre des opérations d'aménagement et de construction.

Madame la sénatrice Monsieur le Sénateur, créer une véritable inégalité entre les secteurs et en contres entre les contribuables, ce qui ne me paraît pas souhaitable du tout, je rappelle que le conseil constitutionnel est particulièrement attaché au principe de l'égalité devant l'impôt. je ne suis pas sûr que la modulation du taux de la taxe d'aménagement, soit le meilleur outil pour promouvoir l'installation d'activités commerciales dans les centre-villes je pense au contraire qu'il vaudrait mieux favoriser par d'autres dispositifs de soutien aux entreprises, notamment aux petites ou moyennes, dans le cadre des politiques de soutien aux outils par les outils économiques des métropoles de la région et parfois l'accompagnement des collectivités, je pense que c'est plus par ce dispositif, que par la modulation de la taxe d'aménagement sectoriels dans des périmètres finalement ça rajouterait en plus beaucoup de complexité. Je vais mettre aux voix, ces 2 amendements identiques, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Ils ne sont pas adoptés, je vais mettre aux voix l'article 43, quels sont ceux qui sont pour, quels sont ceux qui sont contre l'article 43 est adopté. 2 amendements identiques, le 13 99, il n'est pas soutenu le 14 62, monsieur l'a menée. Merci, merci, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, donc à l'initiative de notre collègue Serge Babary, cet amendement vise à insérer un article additionnel au niveau du code général des collectivités territoriales, il rappelle que la taxe locale sur la publicité extérieure a remplacé la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes ce produit de TLPE est devenue d'une certaine manière, très dynamique, mais malheureusement, comme ça a été répété de nombreuses fois les entreprises vivent actuellement une crise sanitaire sans précédent. Donc de suite une suppression de de cette taxe T. L. T. L. P. E. constituerait une aide importante pour les commerces de proximité qui ont plus que jamais besoin d'un accompagnement certes la TLPE est une taxe facultative et les communes qui l'ont institué sont aujourd'hui confrontées à une baisse importante de leurs recettes : une augmentation de leurs charges de ce fait, ne peuvent plus se permettent de la supprimer ainsi si le présent amendement on propose la suppression, il prévoit que cette perte de recettes seraient compensées par l'État via une majoration de la DGF. De ce fait, la suppression de la TLPE s'inscrit par ailleurs dans l'objectif du gouvernement qui vise à réduire la pression fiscale des entreprises donc de défendent le monde économique, telle est l'objet de cet amendement. Avis de la commission. Un avis défavorable, ce n'est pas une surprise parce que il y a, c'est une suppression qui est proposé, alors, on connaît la difficulté de la TLPE il est possible de faire des oeufs amendement ou des réductions actuellement d'ailleurs un certain nombre de collectivités, il procède mais là le dispositif telle qu'il est prévu, selon moi, il ne marche pas puisque, il y a pas de modalités de compensation de cette ressource fiscale du bloc communal donc vraiment une demande un avis défavorable.

je crois que suscitait samedi, ou vendredi les taxes funéraires sont passés à la trappe, enfin on peut supprimer toutes les taxes qui alimentent les Budgets communaux et puis espérer une compensation au travers de la DGF, franchement, on sait ce qu'il en est, donc ça me semble d'une, ça me

utilisent des moyens qui, qui franchement détériore largement les les paysages, donc elle a un double objectif : cette taxe et et je pense qu'il est tout à fait judicieux de la préserver, telle qu'elle est. Monsieur le écoutez, compte tenu des explications du rapporteur général, monsieur le ministre je, moi je, je retire cet amendement. Je vais mettre aux voix l'article 43 bis, quels sont ceux qui sont pour, quels sont ceux qui sont contre lui s'abstiennent il est adopté, je mets aux voix, l'article 43 terre quels sont ceux qui sont en Contre qui s'abstiennent il est adopté. Après l'article 43 terre un amendement 13 38 présenté par Monsieur Capo Canellas. Merci monsieur le président, Monsieur le président Monsieur mes, mes chers collègues, il s'agit d'apporter une précision, s'agissant de la taxe d'aviation civile et de la taxe de solidarité pour les billets d'avion, spéciale de la taxe, pardon de l'aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, ces tarifs sont différenciées en fonction de la zone de destination finale du passager, en l'occurrence un tarif minoré s'applique lorsque la destination finale est situé dans la zone constitue bien sûr par la France, mais aussi les autres États membres de l'Union européenne et enfin les autres et les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse un tarif normal, par contre, applique lorsque sa destination finale se situe dans la zone constituée par les autres États l'ajout dans le périmètre de la zone géopolitique européenne un critère géographique à savoir un État situé à moins de 1000 kilomètres de la France continentale a pour objectif principal de se rapprocher des systèmes des des autres pays européens qui, eux, disposent d'une taxe sur les billets d'avion dont les tarifs sont définis selon une liste nominative de pays par exemple pour l'Allemagne, ou bien qui sont définis selon un critère de distance, comme l'Autriche et la Suède, donc voilà l'objet de cet amendement. Avis de la commission. Je sollicite l'avis du Gouvernement sur cet amendement, qui ajoute : finalement à critère géographique dans le périmètre de la zone géopolitique européenne pour laquelle il y aurait ou Avis du gouvernement. Merci monsieur le président, comme l'a dit monsieur le sénateur, ça permet d'apporter une précision utile dans le cadre de la convergence européenne, donc l'avis est favorable. Je mets aux voix cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, l'amendement est adopté. Un amendement 13 39 Monsieur Capo Canellas. Merci monsieur le président, il s'agit. Cette fois, de, d'une précision s'agissant de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, nous avons pour la loi de finances 2020 largement réformer cette taxe de solidarité, on le sait, dans le sens d'un d'un alourdissement, il s'agit simplement de donner une précision pour l'ensemble des compagnies puisque nous avions conditionné la possibilité de moduler à la baisse pour certaines destinations en à l'accord que la Commission européenne, devait nous donner cet accord n'est toujours pas intervenue donc il s'agit, disposer que pour l'avenir, nous attendons encore que cet accord soit donné avant éventuellement de pouvoir moduler à la baisse, donc voilà, c'est une précision qui va dans le sens de la rigueur. Avis de la commission. Je vais à nouveau sollicité l'avis du gouvernement, puisque à la fin de la défense que vient de faire le questeur Vincent Capo Canellas, s'il a effectivement dit qu'il manquait encore actuellement la vie et surtout l'accord de la Commission européenne, donc si Monsieur le Ministre, vous ne pouvez nous dire où en est l'examen. Merci monsieur le président, la vie est favorable, c'est une clarification et qui est utile et elle sécurise l'application d'un dispositif fiscal par une prise de position formelle de la commission qui le valide donc c'est c'est favorable et c'est une pression qui effectivement bienvenue. Je mettre au revoir monsieur le rapporteur. Quels sont ceux qui sont pour. Contre : ils s'abstiennent adopté. Un amendement en 75 Monsieur Jacquin. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, chers collègues, cet amendement vise à proposer de tenir en compte de l'aspect extrêmement polluants, des navires de croisière, particulièrement lors de leur stationnement dans les ports alors comme à chaque fois on nous dit qu'il faudrait un dispositif international international éventuellement de taxation, cet amendement, vous propose de mettre en place un dispositif qui ressemble à la taxe de séjour pour le tourisme appliquées aux navires de croisière lorsqu'il séjourne dans un port français, l'association très fiable, qui s'appelle Transport et Environnement a démontré le pouvoir considérablement polluants de c'est fioul lourd maltraités et donc envoyer un signal aux compagnies de croisière nous semble être un dispositif intéressant, j'ai bien dit un signal ça ne mettra pas mal l'activité qui est en ce moment très affecté, j'en conviens mais on regarde plus loin que la situation d'aujourd'hui, je vous remercie, C'est effectivement finalement tout le paradoxe, parfois des des amendements qui. Sont confrontés à une une intention louable de travailler à réduire notamment la pollution atmosphérique, là en l'occurrence des bateaux de croisière d'avoir dans la situation actuelle, finalement est-ce que on n'appuieraient pas là où il y a déjà de la difficulté puisque c'est des compagnies qui ne ne ne ne réalise plus de chiffre d'affaires, deuxièmement derrière quand même, on s'aperçoit là aussi parfois de de de la contradiction dans la demande des uns ou des autres, c'est le fait que ça crée une enfin une valeur ajoutée sur le la vitalité économique des territoires où se trouve c'est c'est un port pour les navires de croisière et troisièmement, je pense que le plus important c'est la mutation à laquelle cette industrie est en train de procéder sur la manière dont

à mon avis, on ne peut pas ne pas la mener avec les acteurs portuaire aérien ou automobile, le gouvernement est défavorable aux augmentations de taxes et, qui plus est, mais, Monsieur le Sénateur, l'a dit, dans une période où tels ou tels secteurs rend compte des difficultés particulières donc même s'il y a une application qui est différée dans le temps, nous considérons que le signal serait par trop négatif que de laisser entendre un secteur que dès lors qu'il sortira la tête de l'eau, il aurait une taxe à quitter immédiatement donc l'avis sera défavorable sur tous les amendements proposant des taxes nouvelles. je vais le retirer parce que je leur mettrais certainement dans le texte à venir, nous dit-on, sur la les propositions climat autour de la Convention citoyenne, j'ai apprécié les argumentaires, je sais, monsieur le rapporteur, sensible aux problèmes de qualité qualité de l'air, je le ramènerai cet amendement parce que le souffrait extrêmement toxique et il faut vraiment vraiment accompagner ses activités de de tourisme non n'essentiel mais importante au niveau économique, je le retire parce qu'effectivement, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est un le signal est pas forcément limpide, il sera plus intéressant de le regrouper dans un texte qui traite du problème climatique et quant à ce que me dit : Monsieur le Ministre, sur le fait que il n'est pas sans si il ne souhaite pas les taxes qui vont sur les carburants, là je crois qu'on a une vraie difficulté, si on veut imaginer un report modal et des évolutions, il faudra forcément discriminer certains carburants par rapport à d'autres, je vous remercie. Les 146 rectifié monsieur oui. Merci Monsieur le Président, cet amendement précise que depuis la loi de finances 2000 19 au niveau de l'IFER, il y a une répartition à 80 % pour les communautés et à 20 % pour les communes, sur les éoliennes et on comprend bien, parce que l'acceptabilité des éoliennes et parfois contesté et donc cet amendement propose d'adopter la même répartition pour ce qui concerne les installations photovoltaïques car on voit bien que là aussi il y a parfois de l'hostilité localement et il importe que la commune soit la plus impliquée possibles pour développer les installations de photovoltaïque parce qu'on le sait, on le sait tous, la, la, le nez, la nécessité de développer les la production d'énergie renouvelable est un impératif important pour notre pays et donc il convient d'encourager l'ensemble des acteurs dans ce sens et et de mobiliser les communes autour de cet objectif c'est le c'est le sens de cet amendement de bon sens.

fait c'est un peu sur le modèle, vous l'avez rappelé de ce qui existe pour lui faire éolien, ceci étant, je ne pense pas qu'il faille amener cette réflexion au détour d'un amendement parce que l'appropriation et surtout l'appréhension globale n'est pas n'a pas été fait et je pense qu'il faudrait surtout peut-être le le présenter une prochaine fois, mais à avoir un diagnostic des d'un certain nombre de situations locales parce que tout dépend par exemple entre la commune, elle intercomités je pense que c'est pas la même chose quand on est peut-être à 20 ou 30 kilomètres d'une agglomération, voire d'une métropole ou quand, dans des territoires à dominante rurale, parfois même en zone de montagne et donc je de mon point de vue cette des éléments qui doivent être pris en compte dans la réflexion pour essayer de trouver le meilleur équilibre effectivement pour permettre que les communes n'aient pas à subir parfois un certain nombre, parce qu'il y a toujours des contraintes sans avoir un minimum de retour et puis être attentif au fait que l'intercommunalité soit aussi porteuse parce que cette le rayonnement ils bénéficient souvent aussi au territoire de cette ou de ces intercommunalités parce qu'il peut aussi y avoir de l'Inter territorialité donc une demande de retrait. Merci monsieur le président sur les questions relatives à l'hiver, je partage ce que dit monsieur le rapporteur, la nécessité qu'il y a peut-être plus de travaux préalables avant de procéder à telle ou telle modification, c'est le cas de l'amendement du sénateur, c'est le cas d'amendements qui viennent ensuite, dans la discussion et parce que ces travaux n'ont pas été menée, il nous paraît aujourd'hui un peu prématuré de modifier les règles relatives à l'hiver, c'est la raison pour laquelle l'avis sera défavorable pour cette seule raison sur tous les amendements relatifs à l'hiver. Oui, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je ne pas rapporteur général, je ne peux pas être d'accord du tout avec les observations et les arguments qui viennent d'être développés. On parle bien d'un surcroît de richesses générées par de nouvelles installations, donc de la richesse supplémentaire, pourquoi est ce que toute la richesse supplémentaire créé irait systématiquement le PCI, est ce que on ne peut pas partager une partie de la richesse supplémentaire qui est créé avec les communes, une toute petite partie c'est un 5ème et on parle bien de la richesse supplémentaire, donc moi je veux bien qu'on aille demander des études d'impact mais ça ça ça n'a aucun sens d'allégement des études d'impact sur des projets à venir, hein, puisque on ne peut pas anticiper les projets à venir, c'est à l'avenir, je dois dire bah si il y a 10000 euros diffère qui est produit la richesse supplémentaire, il y a 8000 qui iront dans les caisses de la communauté et 2000 qui rentre dans les caisses des communes de la commune concernée mais c'est de bon sens. Je vais donc mettre aux voix, cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont compte. Qui s'abstiennent.

Quels sont ceux qui sont contre. Ils sont adoptés. 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune mais ils ne sont pas soutenus. Donc à l'article que 43 terre un amendement 12 63 Madame très ville. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en matière de production énergétique, la fiscalité actuelle est à rebours les objectifs que nous nous sommes fixés, particulièrement en ce qui concerne le soutien à l'hydroélectricité, la filière hydroélectrique représente la 2ème source d'énergie française elle totalise 12 % de la production électrique totale et 49 %, de l'énergie renouvelable produite en 2018 faisant donc de cette énergie la première source d'énergie renouvelable en France

l'hydroélectricité est ainsi électricité la plus propre en matière d'émissions de gaz à effet de serre, les unités de production électrique sont aujourd'hui soumises en termes d'impôts Directs à l'impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l'IFER, une centrale électrique est imposable à lui faire à partir d'un seuil de puissance électrique installée ce seuil varie en fonction du type de centrale concernées et pour les centrales hydroélectriques éoliennes et photovoltaïques, ce seuil est de 100 kilowatts de puissance installée un seuil, vous en vous en conviendrez, relativement faible, à contrario, les centrales thermiques sont quant à elles, imposées au titre de l'hiver, à partir d'une puissance de 50 mégawatts de puissance installée face à cette situation, l'ensemble des acteurs de la filière hydroélectrique sont son est unanime : il souhaite reprendre les droits fondée en titre et pouvoir réhabiliter les moulins à l'arrêt, cependant, il se heurte à une fiscalité en vigueur qui représentent un réel frein au développement du secteur, cette énergie hydroélectrique est la plus rentable, pourtant en matière énergétique, comme le montre le facteur de charge plus la valeur du facteur de charge est élevé, plus l'installation considérée s'approche de sa capacité de production maximale

que représente cette petite hydroélectricité, elle ne nécessite ni retenue ni vidange ponctuels susceptibles de perdus de perturber l'hydrologie, la biologie ou la qualité de l'eau, elle présente un bilan écologique donc positif non seulement en ne perturbant pas les écosystèmes mais en permettant à l'entretien des cours d'eau, ces petites centrales évitent ainsi les principaux inconvénients des centrales hydroélectriques traditionnelles, c'est pourquoi nous devons encourager leur développement, la seconde caractéristique de la petite hydroélectricité réside dans le fait que celle-ci est composée principalement de centrales dites au fil de l'eau E fonctionne donc continuellement et forment un apport stable en énergie et assure, vous le savez aussi la stabilité du réseau lui-même, c'est pourquoi le présent amendement propose de : d'une part, de relever le seuil d'assujettissement à les faire pour ne plus imposer les petites centrales et relancer l'investissement, d'autre part, modifier l'imposition des transformateurs en distinguant la production d'électricité verte électricité ici issues de combustibles fossiles au moyen d'une diminution de l'hiver pour les usines de production d'électricité verte. Ce sera une demande de retrait, madame la sénatrice pour votre amendement qui provoquerait vous l'avait pas dit mais c'est bien sous-entendu une baisse de recettes non compensés significative pour les collectivités territoriales d'implantation de des centrales hydroélectriques pour tout vous dire, j'entends l'argumentation vous développer, je souscris au fait que, on devrait d'abord d'abord retravaillé parce que il y a plusieurs plusieurs étapes et plusieurs étages dans votre réforme, et là encore, je ne suis pas sûr que ce soit au travers d'un an d'un simple amendement ou d'un amendement en PLF que nous pouvons, et que nous devons procéder à ce type de modification mais le le sujet et la manière dont vous l'abordez, je pense, doit nous interroger et nous intéresse mais malgré, malgré tout ça, une demande de retrait. donc je suis bien d'accord

Sur le président seul ministre, chers collègues, cet amendement proposé par notre collègue Gremillet a pour objet de permettent aux collectivités territoriales qui le souhaitent d'exonérer d'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux, les stations de transfert d'énergie par pompage l'énergie hydroélectrique dans tous ses usages devant être promu. C'est un avis de sagesse qui se justifie à la fois par l'objet une possibilité d'exonération facultative et par, finalement c'est nous l'adoptons depuis plusieurs années dans le cadre de l'examen du PLF. Je mettre aux voix, pas maintenant, qui a reçu un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du Gouvernement quels sont ceux qui sont en Quels sont ceux qui sont contre, ils s'abstiennent adopté. Le 13 92 Madame Schillinger pas soutenu. Un article 10 84 de Madame Sollogoub Monsieur Delcroix Obama. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, cet amendement vise à favoriser le développement des énergies renouvelables, par le biais de la petite hydroélectricité, ils proposent donc de permettre aux départements, aux communes ou aux EPCI à fiscalité propre évidemment si ces collectivités le souhaitent d'exonérer temporairement pour la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments affectés à la production d'hydroélectricité je redis bien si ces collectivités, de fait, il s'agit évidemment pas d'en d'en faire une obligation. Un avis de sagesse, ça a bien été rappelé par Bernard Delcros, c'est sur la base du volontariat. Donc selon moi le le l'amendement mérite effectivement non seulement notre attention, mais davantage sûrement notre soutien. Le gouvernement. Je vais mettre aux voix, quels sont ceux qui sont pour. Ils sont contre, qui s'abstiennent, qu'il est adopté. Le

bonjour monsieur le président, Monsieur le Ministre, mais mes chers collègues, il s'agit malheureusement d'une petite taxe qu'on vous propose de mètres sur les surfaces de stationnement comme des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce sur une surface de vente de plus de 2500 mètres carrés donc ça vous donne quand même l'an l'ampleur pour vous dire que ça a été mis en oeuvre en 2015 par la seule région Île-de-France cette taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement annexé aux locaux à usage de bureaux locaux commerciaux locaux de stockage a permis de financer des dépenses d'investissement de la région Île-de-France en faveur des transports en commun, donc cet amendement il proposerait d'étendre à l'ensemble du pays, ce principe, afin d'apporter une une contribution importante au budget de l'actif et au développement d'investissement donc pour une mobilité vertueuse tout à l'heure, on a eu l'artifice, l'artificialisation des sols mais on a aussi besoin de développer les, les, les transports en commun et des circulations douces, merci. Avis de la commission. Un avis défavorable, monsieur le sénateur, je rappelle que nous avons adopté, en première partie du PLF, une hausse de 400 millions d'euros d'euros du produit de la TICPE, affectée à l'AFITF en 2021 et que les ressources de cette agence pour 2022 seront fixés dans le prochain projet de loi de finances.

et juste pour rappeler que dans un certain nombre de cas, ce sont les collectivités qui finissent par payer cette taxe, soit parce qu'elles ont le Parking en régie, soit parce que dans le contrat de délégation ou de concession, cette clause force majeure se répercute directement sur les collectivités d'élégantes, donc je ont finalement on frais payés par les collectivités, cette taxe, donc je pense que c'est pas très heureux, comme la taxe qui en Île-de-France n'est pas très heureuse non plus. je fait maintenir l'amendement puis en temps voulu Madame Lavarde nous donnera des exemples concrets, parce que c'est, c'est bien d'avoir une réponse globalisante mais nous donnera les collectivités en cause. Donc je mets aux voix cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre ou s'abstiennent, elle n'est pas adopté. L'article 43 terre toujours 428 rectifié. Madame Paoli-Gagin. Oui, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, il s'agit d'un amendement qui propose de revenir sur une expérimentation de 5 ans maximum d'une éco-taxe pour les véhicules de plus de 3 tonnes 5 qui empruntent les voies ou portions de voies de circulation dite voie rapide, la mise en place de cette écotaxe serait laissé à la libre appréciation des départements, l'objet de cet amendement, c'est de répondre aux problèmes des départements qui subissent un trafic routier extrêmement important, un trafic excessif de poids lourds qui crée des problèmes environnementaux de santé publique, de vie quotidienne très importants pour les populations, il convient de tenter d'y remédier en tentant l'expérimentation volontaire d'une écotaxe. Alors cet amendement soulève un problème d'importance : la contribution des poids lourds qui traversent. qui utilisent les infrastructures routières ou autoroutières sans eux, notamment étrangers, sans eux, apporté aucune contribution. Je rappelle que ce sujet, il a fait un peu de dégâts dans l'opinion, dans un 1er temps avec des bonnets rouges puis avec des gilets jaunes, je ne sais pas si vous cherchez si on cherche à travers ce cet amendement d'appel, de faire de l'orangé, mais en tous les cas je je ne souscris pas voilà à ce à cet éventuel changement de couleur sur un sujet. Pour lequel, néanmoins, le gouvernement avait annoncé il y a 2 ans, vouloir travailler avec l'ensemble des parties prenantes, parce que ça reste un sujet particulièrement complexe, je ne pense pas, néanmoins, que la manière dont eux par cet amendement, vous proposez de revenir sur le dispositif en alors je pense que c'est plutôt un amendement d'appel mais en requérant une taxe départementale soit la bonne solution et surtout au bon moment pour les raisons que j'ai évoquée, d'où la demande de retrait. Je vais mettre aux voix, quels sont ceux qui sont pour. Qui s'abstiennent pas adopté. Il y avait, merci monsieur le président, donc, cet amendement vise à rendre obligatoire pour l'employeur, l'administration employeur la prise en charge d'un forfait mobilité durable destiné aux salariés. Le dispositif du forfait mobilité durable mis en place en 2019 par là l'homme. Repose actuellement sur le volontariat de l'employeur, son déploiement reste donc très limitée, d'ailleurs, l'Ademe avait constaté en 2018 seuls 237000 salariés soit moi, soit moins d'1 % de la population actif bénéficier de ce dispositif, qui à l'époque s'appelait l'indemnité kilométrique vélo le rendre obligatoire, et donc l'étendre à une population plus large c'est tout cet outil permettrait pourtant de modifier profondément les modalités de déplacement au sein des entreprises ou des administrations en incitant la pratique des modes de transports doux ou du covoiturage. Je pense qu'on ne peut que l'encourager dans ce sens. Avis de la commission. Alors, encourager les mobilités douces et l'utilisation du deux-roues non motorisé, donc du vélo, pourquoi pas, par contre je ne souscris pas au caractère obligatoire de ce forfait mobilité durable, je crois que, il faut aussi se dire que dans le contexte actuel, vous voyez bien que cette de, finalement, ce serait des contributions supplémentaires demandés aux entreprises, notamment aux petites et aux moyennes entreprises, raison pour laquelle je un avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement, quels sont ceux qui sont. Pour.

Monsieur le président, monsieur le ministre, cet amendement proposé par notre collègue Bormio Fontan entend exonérer les SDIS de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, énergétiques, en effet, certaines professions sont déjà exonérés en tout ou partie de la TICPE, comme par exemple les taxis ou les transporteurs routiers, le SDIS en sont redevables de plein droit, alors même que qu'une directive du 27 octobre 2003 rend possible une exonération partielle pour les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers, y compris des taxis, la collecte de déchets des forces armées et l'administration publique, les personnes handicapées, les ambulances, il faut constater qu'en zone rurale, le manque de prestataires privés, ce qu'on appelle les carences ambulancière amène bien souvent les sapeurs-pompiers à prendre en charge le transport sanitaire dit non urgents le remboursement au SDIS de leurs frais d'intervention pour carence ambulancière effectif s'effectue sur la base d'un forfait de 118 euros très largement inférieur au coût réel de la prestation qu'on peut évaluer à 190 euros d'ailleurs, c'est toujours aussi extrêmement compliqué des fois d'aller qualifier les carences ambulancière entre le SDIS le SAMU pour le remboursement, c'est donc un coût qui pèsent de façon importante sur les finances qui sont déjà fortement contraintes des collectivités territoriales, je rappelle d'ailleurs que ce sont les conseils départementaux qui sont le curseur d'ajustement des coûts supplémentaires des finances du SDIS et notamment récemment, le gouvernement a décidé l'augmentation de la prime de feu qui n'a pas cette 19 à 25 qui a un coût global de l'ordre de 80 millions d'euros, qui n'est compensée que partiellement, à hauteur d'une petite moitié entre 30 et 40 millions d'euros par la suppression de la surcotisation employeur à la scène se serait donc le une décision bienvenue que d'exonérer le SDIS de cette taxe, qui pourront alors utiliser ces nouvelles ressources financières pour compenser une partie de l'augmentation des charges décidées par l'État ou alors continuer leurs efforts d'investissement qui sont liés aux nouveaux risques, merci. C'est le sénateur Vogel, je comprends, et notamment l'aspect plus particulier sur les services d'incendie et de secours qui est finalement un peu la fragilité du dispositif dans où il n'y a pas possibilité d'accéder à votre demande, en raison d'une contrainte européenne d'ailleurs le ministre, il y avait déjà répondu, en 2018 et ça n'a pas changé depuis le problème de la carence ambulancière, là on voit qu'il a, il y a, c'est là où je pense, il y a un sujet est ce qui doit être est ce qu'il doit y être répondu par l'exonération telle que vous la proposer, je pense que non, mais en vous disant non je n'offre pas non plus la solution à tous les cas que vous évoquez, moi je pense qu'il nous faut être en adéquation avec le droit européen et je pense enfin qu'il faut peut-être aussi être attentif à ne pas multiplier les cas d'exonération de la TICPE, c'est-à-dire on ne pourrait pas le faire non plus pour et il y aurait pas de raison pour l'ensemble des administrations publiques. Du gouvernement. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur souligne que j'avais fait cette réponse en 2018, je l'ai fait, en 2009, je l'ai fait, en 2020 sur les différents pays, les faire comme en première partie de ce PLF c'est un état de fait liés au droit européen qui nous empêche de donner une réponse favorable à ce type d'amendement l'application concernerait tous les services publics ou où aucun, en dehors de ce précisément listés par la directive, c'est la seule raison pour laquelle, de manière constante, l'avis est défavorable. Je vais retirer cet amendement mais ce que j'aimerais, c'est que vous nous fassiez une promesse, c'est de revoir ces problématiques d'indemnisation des carences ambulancière privé parce que ça pèse extrêmement sur le coût des SDIS, par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie difficulté de détermination de la carence ambulancière privé pour un certain nombre de raisons, et souvent des raisons budgétaires au niveau des SAMU qui n'ont pas assez de finances pour indemniser les carences ambulancière et en fait ça vise à reporter des Budgets d'État sur les Budgets des conseils départementaux en refusant d'indemniser les coûts réels des carences ambulancière donc je retire cet amendement mais Monsieur le Ministre, j'aimerais bien que vous puissiez nous indiquer que vous avez vous occuper de façon sérieuse de ce sujet-là Olivier Richefou d'ailleurs, le président de la CNIL l'a relevé à plusieurs, à plusieurs cas et je souhaiterais que vous pouvez vous puissiez vous exprimerez très rapidement sur ce sujet, merci.

j'aimerais, monsieur le Ministre que auprès de vos collègues, à la fois du ministre de la Santé et de l'Intérieur, il y a eu une proposition de l'association des départements de France, qui propose ce remboursement à hauteur de 251 euros aujourd'hui, ça se trouve être entre 2 sont 18 enfin 100 118 124 euros il y a eu des propositions de faites, il y a eu 2 rapports qui ont été rendus par l'inspection générale de l'administration et des affaires sociales sur ce sujet, il est vraiment urgent maintenant de de décider la balle est dans le camp du gouvernement, il faut qu'ils décident de l'indemnisation de cette situation, c'est quand même par ricochet aussi la situation de la désertification médicale et il faut aujourd'hui que les départements souhaite accompagner parce que en effet de plus en plus, les indices sont amenés à un ça intervenir sur des opérations non prioritaires et de surcroît ça a pour conséquence un de de ne plus dynamiser le bénévolat, et d'autre part, les employeurs sont de plus en plus hésitants à avoir des sapeurs-pompiers volontaires, parce qu'il les voyait partir sur des opérations non prioritaires, donc vraiment il revient maintenant au gouvernement en responsabilité de prendre cette décision pour mettre fin à cette situation. C'est le ministre. Un mot pour dire un petit peu, madame la sénatrice, que je ne portais pas de promesses que je ne sais pas tenir que cela relève d'autres champs ministériels et que je ne suis pas au fait des discussions il y a un second par Monsieur Vogel pour lui dire que je n'ai pas besoin ni d'injonction, ni de ton véhément pour m'occuper des choses sérieusement, comme vous l'avez évoqué.

monsieur Kahn. Président, monsieur le ministre, ce rapporteur général, chers collègues, c'est un amendement d'appel de notre collègue Claude Kern, qui vise à proposer à ce que, d'ici le 1er juillet prochain une loi quinquennale des finances définissant les objectifs et les priorités de la fiscalité écologique et je dirais le le les tendances de la fiscalité écologique sur la période quinquennale puisse être adopté, donc c'est un amendement d'appel, il est important que l'on sache vers où on va. Avis de la commission. l'affectation des recettes relève de ce qu'on est en train de faire des lois de finances, je pense que dans l'objet, il faut être attentif à ne pas, comment dirais-je, à ne pas par trop se divertir, raison pour laquelle je suis j'émets un avis défavorable. Avis du gouvernement.

Merci monsieur le président, il s'agit d'un amendement de mon collègue, Emmanuel Capus, vous le savez, la suppression du compte d'affectation spéciale Transition énergétique a été après de longs débats, voté en loi de finances pour 2020 acte a été pris de cette suppression, malgré les nombreuses questions qui demeurent temps suspens dans sa note d'analyse de l'exécution budgétaire 2019 relative au CAS Transition énergétique, la Cour des comptes, rappelle que la Caisse des dépôts et consignations gère le fonds casse la Cour demande à ce que soit réalisée avant le 30 juin 2021 une évaluation détaillée des coûts et des économies engendrées par cette reprise en interne, l'amendement que proposée par mon collègue vise à reprend de la recommandation de la Cour des comptes, en demandant au gouvernement un rapport présentant une évaluation détaillée des coûts et des économies engendrées par une telle reprise en interne.

Merci monsieur le président, le gouvernement a lancé en février 2020, un appel à manifestation d'intérêt pour les projets de création d'unités de production de biocarburants de 2ème génération pouvant être utilisés dans le secteur aéronautique, c'est une excellente chose, cet appel à manifestation d'intérêt s'inscrit dans le cas de la feuille de route nationale pour le déploiement des biocarburant aéronautique durable, on voit à ce stade que la mise en place d'une telle filière apparaît complexe, or l'article 15 du projet de loi de finances prévoit une extension de la terrible au secteur aérien qui entrera en application au 1er janvier 2022, donc on a une difficulté entre l'horizon 2022 pour la Syrie et l'horizon 2024 qui semblerait apparaître dans le cadre, cet appel à manifestation d'intérêt le présent amendement pose ce ce problème de temporalité, et propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants, ce rapport devra permettent d'apprécier la cohérence entre la date d'application de la par rapport à l'émergence effectif d'une production de biocarburants sur le territoire national et d'envisager la question de l'adapter. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en effet, le l'amendement est identique : il vient d'être excellemment défendu par notre collègue de quoi s'agit il s'agit essentiellement de vérifier qu'au moment de l'entrée en vigueur de cette taxe qui vise à inciter l'incorporation de biocarburants dans l'aviation, au 1er janvier 2022, c'est-à-dire demain, il y a sur le marché des carburants qui permettent d'échapper à la taxe, en effet, puisque celle-ci vise à encourager l'utilisation des biocarburants donc cette vérification et au moins légitime, avant qu'on applique la taxe sinon c'est plus une taxe d'incitation, c'est encore une fois, une taxe de rendement, donc je vous invite aussi très vivement, mes chers collègues, à à voter pour une fois, cette demande de rapport, même si vous connaissez la répugnance traditionnelle, la commission des finances à cet égard.

j'avais l'occasion d'auditionner les dirigeants, par exemple, d'Air France, mais effectivement dans le cas de la discussion du du PLF nous avons souligné la difficulté peut-être d'être parfaitement au rendez-vous en 2022 sur le sujet des biocarburants pour le secteur aéronautique et je pense que ce sujet d'ailleurs, il faut aller faut aller au bout de la réflexion et du diagnostic, c'est dans les biocarburants, quels types de biocarburants mobilisant, on va dire qui quelle quelle production parce que cette, ce sera aussi un enjeu d'aucuns le font entre le le la question de la production de de ressources végétales et puis certains sujets autour de l'alimentation, donc d'éclairer les horizons différents, pour reprendre les les mots du Sénateur Capo Canellas, ça me paraît une décision en tous les cas, a encouragé et qui doit aussi nous permettre ensuite de pouvoir nous prononcer en meilleure et j'espère en toute connaissance de cause. Comme sur toutes les demandes de rapport défavorable monsieur Bazin. Oui merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, juste à un mot très rapidement complémentaires ce qui a pu être dit dans le débat, jusque là, c'est que, au 1er janvier 2022, c'est peut-être pas la période la plus intéressante pour pénaliser davantage Air France qui va avoir de redoutables défis à relever dans les années qui viennent, ce souvenir également que les avions des compagnies étrangères notamment peuvent faire le plein ailleurs que sur le territoire national pour venir concurrencer très défavorablement notre compagnie nationale, nous prenons aussi les intérêts d'Air France à coeur dans cette affaire. Oui, monsieur le président, d'abord, mon collègue Bazin a très bien dit que pour une fois et je remercie le rapporteur général en fait une exception à la règle concernant les les rapports mais qu'est ce qu'on veut dire simplement ici, c'est qu'il faut une filière de biocarburants et ça nous paraît la première étape vers une transition écologique plus forte du secteur aéronautique, on sait qu'après on ira sans doute vers l'hydrogène et que ça réclame là aussi en saut technologique dans cette première étape nous paraît indispensable, voilà, pour autant, on dit qu'il ne faut pas forcément taxés avant que la filière de biocarburants existe et il semble que l'appel à manifestation d'intérêt que le gouvernement a lui-même réalisé conclu à ce que la filière ne sera pas présente avant 2024 d'où on pose la question : est ce qu'on peut avoir la terribles avant alors que la filière n'existe pas. C'est pas cher, oui merci monsieur. Le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au moment où l'État, selon la presse qui est mieux informée que le Parlement devrait investir dans Air France, entre 4 à 7 milliards d'euros. Il serait peut-être bon effectivement que tout soit présent et à l'oeuvre et vous comprendrez que ce rapport et c'est après moi assez utile certes à titre exceptionnel, parce que ça a pas vraiment de sens qu'on fasse injonction mais là, monsieur le ministre. Si vous pouviez aussi nous éclairer sur cette petite dépense certes pas budgétaires à ce stade, ça va être du capital, enfin c'est quand même assez paradoxal qu'on appelle les choses par la presse, à ce niveau-là. Je vais mettre aux voix, cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, ils sont adoptés. l'article car 43 ter toujours un amendement 105 monsieur Capo Canellas. Merci Monsieur le Président, cet amendement concerne la mise en oeuvre d'une taxation environnementale du secteur aérien au niveau international, ou à défaut au niveau européen, on sait que beaucoup convergent dans cette cette direction-là et il s'agit de regarder ou est-ce que nous en sommes aujourd'hui puisque les discussions sont à à l'oeuvre au niveau de l'Union européenne sur une possible taxation du kérosène ou sur une réforme du système d'échange des quotas d'émissions visant donc à diminuer le nombre de quotas alloués gratuitement et il nous semble, c'est effectivement au niveau européen, que la discussion doit avoir lieu, je crois que c'est une bonne chose dans ce contexte, le présent amendement prévoit que le gouvernement remettra alors je suis désolé, c'est là aussi un rapport mais il y a pas d'autre façon de faire non seulement un rapport avec une une information exhaustive sur les projets de taxation du transport aérien au niveau international ou européen pour voir où est-ce qu'on en est pour avancer dans cette direction-là mais également envisager les solutions qui. Pourrait être mis en oeuvre pour concilier à cette éventuelle taxation européenne avec celle que nous venons de mettre en place, s'agissant de la taxe de solidarité sur les billets d'avion parce qu'il faudra aussi à à ce moment-là, se poser la question de la conciliation des 2 systèmes. Et de la Commission. Ce sera un avis de sagesse de la même manière que les années précédentes, puisque l'an passé déjà, nous avons, nous avions pardon adopté cet amendement. Avis de du gouvernement.

qui sont à même de délivrer des rapports, la commission des Finances peut demander via l'article 58 de des rapports à la Cour des comptes, il y a tous les rapports d'inspection générale interne, il y a des rapports d'organismes divers bien sur les 500 km/s, mais aussi des organismes associés à l'État ou au gouvernement, France Stratégie et autres je pense que de temps en temps, devra avoir un système lorsque nous avons des amendements de demandes de rapport où on pourrait transférer cet amendement à telle ou telle commission pour voir si un rapport existe, si une demande de rapport est en cours, ou si le Sénat pourrait formuler une demande de de rapport, ce qui ne joue vite ils éviteraient de nous tourner systématiquement vers le gouvernement pour dire un rapport est plutôt nous aider nous appuyer sur l'existant qui est quand même assez massif en France pour pour évaluer j'ai j'ai cité quelques organismes mais il y en a beaucoup, beaucoup beaucoup d'autres. Une courte réponse Monsieur le Sénateur, d'abord, vous l'avez rappelé : nous ne sommes pas des adeptes à la commission des finances et rends assez peu d'avis favorables, alors parfois je suis battu, enfin, où la Commission est battu, après il faut qu'on fasse la part des choses souvent dans les rapports quand les rapports sont demandés si ça peut être des rapports du gouvernement ou des oeufs différentes institutions organismes qui travaillent en coordination avec le gouvernement, mais parfois c'est aussi pour ce pour essayer d'avoir un un état des lieux où une une expression par par un tiers, voilà donc j'entends bien, je je souscris à votre demande, mais vraiment je je crois pouvoir dire qu'on nous fait plutôt le reproche de voilà de de proposer ou de rendre des avis négatifs pour éviter l'accumulation et pour tout dire je pense parfois, on se fait plaisir, le temps d'une défense d'une proposition et puis après on oublie une partie de la demande en chemin. Au Canada. Oui monsieur, monsieur le président je vais juste insister sur un point, c'est qu'on a en France, le génie de la taxation. Qu'est ce que dit cet cet amendement, il dit simplement que si on pouvait écrire dans la loi que lorsqu'il y aura une taxation européenne sur le kérosène ou sur les émissions du secteur aérien, hé bien à ce moment-là, il faudra qu'on en tire la conséquence sur nos propres taxes nationales et notamment on a créé une taxe additionnelle sur la taxe de solidarité sur les billets d'avion et on est allé en avant par rapport à la négociation européenne, il faudra m'ont donné, se poser la question de l'équilibre général des taxes en France dans ce secteur-là, voilà c'est tout ce que cet amendement dit alors il y a pas d'autre façon de faire que que que la façon qu'il a été utilisé, qui effectivement celle du rapport, mais si on pouvait écrire dans la loi que lorsqu'il y aura une taxation européenne, il faudra adapter la télévision nationale, ça serait encore mieux, ce n'est pas le cas. Je vais donc mettre aux voix, cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont compte. Qui s'abstiennent il est adopté. Je mets aux voix, l'article 43 terre quels sont ceux qui sont pour. Contre qui s'abstiennent il est adopté.

Quels sont ceux qui sont pour. Contre s'abstiennent adopté l'article a supprimé.

Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ne sera pas en général, c'est un amendement qui concerne le crédit d'impôt, audiovisuel, vous savez, la France est un grand pays, culturel et il importe que nous disposions d'outils, nous en avons fiscaux pour cela mais chacun en est bien conscient de la période est particulièrement difficile pour ce qui concerne la production audiovisuelle, par exemple, ce qui était orientée sur les tournages à l'international, il y en a quasiment plus, parce que il n'y a quasiment plus de déplacements et et donc il importe de pouvoir se recentrer sur le national sur le territoire national et en l'occurrence de pouvoir encourager les les productions, vous le voyez bien aussi le contexte fait que ben, il y a beaucoup d'incertitudes beaucoup de de producteurs souhaitent réaliser à minima, un certain nombre de production, donc l'idée de ce cet amendement est simplement de réduire de 2000 euros actuellement, le seuil minimal permettant de bénéficier du crédit d'impôt pour la minute de le réduire à 1500 euros à 1500 euros compte tenu du contexte que nous connaissons de façon à encourager cette production audiovisuelle et ce à partir de 2022, c'est-à-dire pour que les exercices à venir en 2021 puissent le prendre en compte et qu'ils soient effectivement applicables en 2022 ceci permettra, nous l'espérons, de pouvoir encourager la production audiovisuelle, sur l'année qui vient. Merci monsieur le président, oui je veux plaider pour le documentaire français plusieurs amendements utile ont été apportées par le gouvernement. Pour relever le taux du crédit d'impôt pour le documentaire, et par exemple pour l'élargir, élargir ses bénéficiaires aux producteurs de captation de spectacle vivant puisque un pan entier de la production audiovisuelle qui est sinistré en 2020, 2021, qui joue un rôle essentiel cette année pour donner aux Français un accès via le petit écran à des représentations de théâtre, d'opéra de danse auxquels ils ne peuvent plus avoir accès autrement puisqu'elles sont enregistrées sans public, donc voilà. Ce qu'a fait de bien, le gouvernement, cependant il y a un élément technique, je parle pour les spécialistes devraient encore être améliorée, s'agissant du documentaire, parce que le plancher de dépenses permettant d'accéder au crédit d'impôt pour la production documentaire avait été fixé dans le passé, de manière à soutenir les grands documentaires en coproduction internationale dont les Budgets sont élevés, or, en l'absence de marchés internationaux possible et face à une crise des engagements des chaînes étrangères, bien entendu, qui rejoint l'impossibilité d'aller tourner dans le reste du monde, par temps de Covid pour des raisons de restrictions sanitaires au déplacement, le budget moyen des documentaires va chuter en 2021 et ainsi un grand nombre de documentaires ne seront plus aidées parce qu'ils n'atteindront pas ce plancher très élevé actuellement fixé à 2000 euros la minute de dépenses éligibles ainsi pour que le crédit d'impôt pour le documentaire ne manque pas sa cible, il est indispensable de baisser ce plancher à 1500 euros minutes en matière de crédit d'impôt, l'efficacité du dispositif pour cela tenir réellement le financement de la production repose justement sur ces détails plancher de dépenses éligibles assiette Eto le maintien d'un plancher trop élevé viderait en 2021, le dispositif d'une grande part de son efficacité pour le financement de la relance de la production documentaire française dont les qualités sont loués dans le monde entier, en résumé, pour répondre à la crise, documentaire, l'utilisation du levier de financement que constitue le crédit d'impôt n'a jamais été plus adapté, mais il faut pour cela descend le plancher à 1500 euros minutes de dépenses éligibles ce souhait bien sûr est porté par l'ensemble de la chaîne de production document. Terre des réalisateurs français, mais je veux vous convainc Monsieur le Ministre, que ce type de dispositif à son efficacité quand il est millimétrée là il faut l'ajuster. le le crédit d'impôt calculé passe 2150 euros à 1000 400 50 euros par minute produites et livrées je veux également signalé puisque cette dépense fiscale représente en fait 14 7 du coup les documentaire sorti en salles en 2019, c'est pour dire que c'est pas le le facteur essentiel la dépense fiscale d'ailleurs le CNC le reconnaît volontiers, et il existe aussi d'autres dispositifs ou d'autres biais pour apporter le soutien, la raison pour laquelle je demande le retrait. excusez-moi, monsieur le sénateur, a souligné monsieur le rapporteur général, ont rappelé que le gouvernement avait fait soit de son initiative sur l'initiative des parlementaires dans les pays de en matière de crédits d'impôts, et alors même que je dis souvent, et nous disons souvent ne pas être favorable aux dépenses fiscales et que nous considérons qu'un grand nombre de dispositifs de défense fiscal de crédit impôt pour le secteur de la culture sont particulièrement inflationniste, d'une part celui-ci particulièrement mais j'ai eu l'occasion de citer, dispositif qui ont 4 ans vu leur coût multiplie par 2 et demi ou par 3, pour les finances publiques, donc le gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques comme il est défavorable à tous les amendements après le 43 sexy, nous considérons que les mesures qui ont été apportées sont opportunes, mais qui n'est pas nécessaire d'aller. Monsieur Assouline pendant l'explication de vote. Les crédits d'impôt effectivement pour le cinéma, on les a défendus comme parlementaire, il a fallu du temps pour convaincre le gouvernement et Bercy en particulier mais on a gagné et le résultat était le suivant c'est que on a gagné des dizaines de milliers d'emplois qui ont été relocalisés et les rentrées fiscales. En contrepartie de cette regain d'activité ont rapporté plus que ce que ça a coûté en termes de crédits d'impôt, c'est ce que j'appelle le bon ciblage, bien entendu, le crédit d'impôt peut être complètement quelque chose de, de, de, de, d'à côté de la plaque qui produit des effets secondaires, pas voulu. Mais là, ça a marché comme ça. La relocalisation des tournages, par exemple, c'est grâce à ce crédit d'impôt en particulier. Alors sur le documentaire, j'aurais pas dû parce que je reconnais ce qu'a fait le gouvernement, alors on me dit ben ça suffit, puisqu'il a fait beau jeu parce que le problème, ce qu'il a fait, a bien marché, mais là, avec la crise du Covid on tombe au-dessous d'un seuil ou ce qui a été fait ne va plus aider le documentaire comme avant puisque pour atteinte, les 2000 euros minutes ça va évincer ceux qui bénéficiaient jusqu'à présent de cela parce qu'ils seront plus tôt à 1500 euros minutes tout simplement, donc si vous voulez, juge que votre dispositif d'origine soit efficace dans feu contexte il faut baisser le taux, je ne demande pas plus, je demande que les mêmes qui est éligible, soit demain et bon bah vous fermez la porte, mais je vous prie de croire que le documentaire français c'est l'excellence, c'est la qualité, et quand on prétend lutter conter fake News contre le n'importe quoi, hé bien il faut soutenir la qualité.

On va regretter. Quels sont ceux qui sont pour.

Un amendement 644 rectifié madame Darcos. Merci monsieur le Président, j'ai bien entendu le ministre anticiper sur sur tous les amendements que je fais présenté ainsi que mes collègues

vraiment aux abois et donc ce qu'on propose dans les amendements à venir et et notamment la celui-là, qui n'est pas une création de crédit d'impôt et est primordial, j'y associe particulièrement Roger Karoutchi et Catherine Dumas qui voulait aussi déposé le même amendement. Et on ne sommes attendus vraiment partout ce secteur, ce crédit d'impôt sur les dépenses pour les dépenses de production cinématographique est un outil économique qui s'inscrit dans la politique du gouvernement, ils ont incité au tournage des films en France ce que disait notre collègue a souligné, tout en soutenant les industries techniques et l'emploi des techniciens en France, le crédit d'impôt, a fait preuve de sa pertinence en étant reconnu comme efficient et a été amélioré à plusieurs reprises lors des dernières lois de finances, hausse du plafonnement, élargissement des dépenses éligibles, etc, pour s'adapter aux besoins des producteurs d'Oeuvres cinématographiques et retrouver sa pleine activité attractivité territoriale face aux mécanismes fiscaux européens concurrents ainsi sur la période 2015, 2018, le taux de délocalisation des semaines de tournage et passer de 37 à 20 à 20 % et les films à plus gros budget sont intégralement relocaliser 97 % été délocalisée en 2015 par ailleurs le document stratégique, de performances du CN, ces 2018, 2020 montre que la dépense fiscale en faveur du cinéma a été identique entre 2017 et 2019 la prévision de dépenses fiscales pour 2020 étaient même en baisse de 5 % avant même la crise liée au Covid, en parallèle, cette crise du Covid génèrent des surcoûts très significatif pour les producteurs de longs métrages, conséquence d'une part des des lacs décalage des productions et d'autre part, des frais induits, notamment pour le protocole sanitaire très strict qui est mis en place sur les tournages qui peuvent désormais reprendre enfin les chaînes de télévision ont enregistré ces derniers mois une chute inédite de leurs recettes publicitaires, cette baisse du chiffre d'affaires en 2020 devrait diminuer significativement le montant leur obligation d'investissement dans la production cinématographique pour l'année 2021, compte tenu de ce qui précède une augmentation temporaire du taux de crédit d'impôt de 30 à 40 % pour les Oeuvres cinématographiques portant sur les seules dépenses engagées sur les années 2021 pourrait se faire à enveloppe quasi constante sans hausse des dépenses fiscales en faveur du cinéma par rapport aux prévisions et permettent aux producteurs de compenser tant le coût de l'engagement du personnel supplémentaire liée aux mesures suite sanitaire pour les tournages, que la baisse des financements des chaînes de télévision en 2021, telle est l'objet de cet amendement, je vous remercie. Ce sera un avis de sagesse alors effectivement le le ralentissement de la production pourrait inciter à utiliser le biais du crédit d'impôt, hein, pour les tournages afin de de reboosté le dispositif j'attire notre attention sur le fait que le dispositif est tout de même coûteuse puisque s'entraîner une majoration de de la dépense fiscale de près de 40 millions d'euros, mais je note aussi que, quand le plan de relance prévoit plus de 100 millions d'euros pour le cinéma y cette un peu plus de 12 millions d'euros, je dirais seulement qui devrait être consacrée au dispositif pour rattraper le retard pris par la production française, ce qui peut apparaître en dans dans ce cas de figure, donc un avis de sagesse. Oui, un mot, madame, monsieur le président, pardon, pour dire que Madame Marcos a raison, ce n'est pas une création de crédit d'impôt, c'est une augmentation de son taux de de 30 à 40 % c'est un dispositif celui que vous ciblez précisément, dont le coût a augmenté de 50 % entre 2016 et 2018 et pour les raisons évoquées au début de cette série qui sont maintenues pour tous les amendements la vie favorable. le président, Monsieur le Ministre, moi j'entends bien, et dans mon propre rapport à la commission des finances sur l'aide du gouvernement au cinéma à la musique, l'audiovisuel, j'ai déjà dit que vous aviez fait et je le reconnais, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, parce que vous avez pris en compte, effectivement, la crise de 2020, sauf que l'essentiel des efforts, c'est un bilan des pertes de 2020. Et personne ne peut penser que 2021 sera une année normale, personne, je vois que l'épidémie repart, vous ne serez peut-être pas en situation d'ailleurs de déconfiner le 15 décembre je doute que vous au rez, ouvrier l'ensemble des structures culturelles à la fin du mois, en clair, la crise est là et, par conséquent, je pense que tous les secteurs culturels vont être à nouveau très gravement touchés en 2021 et à un moment, il y a, il y a des arbitrages, je, je sais bien que vous avez un endettement considérable un déficit considérable mais comme dirait d'autres je, je vois des des aides à certains secteurs tout à fait utile mais dans le secteur culturel, pardon, Monsieur le Ministre, vous le savez bien, chez les particuliers, c'est peut-être malheureusement, un des premiers secteurs d'arbitrage négatif, ce qui veut dire que forcément ce sont des secteurs qui vont être très gravement crise en 2021 et donc moi j'aurai l'occasion tout à l'heure de défendent rapidement un amendement pour les éditeurs de musique, mais c'est un secteur qui est totalement en crise et les aides 2020 ne suffiront pas pour passer le cap 2021, on vous demande franchement, même si c'est de manière très temporaire de soutenir tout ce secteur culturel 2020, 2021 pour qu'il puisse passer le cap et être avec l'ensemble des Français à la disposition et de de de l'État mais aussi de la culture en elle-même, dès la fin 2021, je l'espère. Madame Dumas. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues, à mon tour je vais apporter évidemment mon soutien à cet amendement, ça a été dit sur d'autres bancs ce crédit d'impôt, on a eu beaucoup de mal à l'avoir maintenant il existe et on a vu qu'il produisait des effets très très positif, notamment sur la délocalisation, ce qu'on vous demande par cet amendement, Monsieur le Ministre, c'est une augmentation temporaire qui concerne l'un de de 2021, alors je serais peut-être moins pessimiste que mon collègue Karoutchi mais on sait très bien que l'année 2021 sera une année très difficile pour la production cinématographique, donc, cet amendement, il répond aux surcoûts importants qui sont du au protocole sanitaire ces surcoûts vont continuer, donc on vous demande pour l'année 2021, de faire un effort, et donc d'accepter cet amendement. monsieur le président, Monsieur le Ministre ne sera pas en général, chers collègues, Catherine Morin-Desailly a préparé un amendement analogues qui auraient pu être en lecture commune effectivement parce que il est important que l'on prenne en compte, comme cela vient d'être évoqué à l'instant, les préoccupations de la production cinématographique française, le contexte, chacun le connaît Catherine du mal, à, à l'instant, vient de l'évoquer, pour ce qui concerne le surcoût des productions du fait des protocoles sanitaires qu'il faut appliquer, mais il ne faut pas oublier non plus que, au plan des télévisions bah les chaînes d'entrée de rentrées publicitaires et donc moins d'argent à consacrée à la production cinématographique et puis et puis regardez la fréquentation des salles de cinéma regardez où est-ce qu'on en est et donc on voit bien que il y aura des difficultés à faire revenir le public dans les salles de cinéma et on espère qu'elle puisse réouvrir le plus rapidement possible, donc il est important que dès à présent, nous prenons les dispositions qui permettent d'encourager une production ce n'est pas de efficiente en France, David Assouline, l'a évoqué tout à l'heure, il faut voir le retour sur investissement que cela génère, on regarde d'un côté le effectivement le coup temporairement, quoi qu'on propose, mais il y a des recettes en contrepartie des recettes de TVA notamment, et on voit bien que plus la production cinématographique française sera excellente est forte et plus le rayonnement culturel de la France à travers le monde s'épanouira également, donc il faut que l'on prenne tout cela en compte. Monsieur Assouline. Oui, là aussi, en effet, les efforts de l'État, grâce aussi à tout ce que l'on a fait au Parlement pour soutenir la filière cinématographique à travers ce levier du crédit d'impôt est à saluer, j'ai hésité sur cet amendement en général parce que je pense que beaucoup a été fait mais le fait que mes collègues qui présente l'amendement disent bien qu'il s'agit de d'une mesure temporaire, c'est-à-dire qu'on ne vient pas encore rajouter à ce qui avait été fait de bien et de suffisant on vient faire en sorte que ceux qui existaient, puisse être maintenue malgré une situation conjoncturelle catastrophique,

parce que c'est l'excellence du cinéma français est quelque chose d'absolument inédit. Par rapport à la taille de la France et même à sa puissance économique, vous avez un cinéma qui écrase tout le cinéma américain, ensuite vous avez un cinéma qui se tient bien mais dans son marché domestique, l'Inde et puis à la France et tous les autres ont pris une baffe se sont écroulés les cinémas classique que vous connaissez, italiens, espagnols, etc, qui ont une renommée qui ont encore des percées ici et là avec des grands réalisateurs mais ces cinémas ont souffert. Pas comme la France, parce qu'à l'un système inédit de financement, et c'est ça concourt au rayonnement de la France de façon incroyable, quand vous allez dans un pays, on vous parle du cinéma français, on vous parle de tels films de tels acteurs et donc je demande que de façon conjoncturelle puisse aider. Avec l'amendement de mes collègues qui vient d'être défendu les les amendements, si on a des similaire, mais si on va celui là, je pense que les autres ont alors personnellement en tous les cas je je voterais pour. Je vais mettre aux voix, ces amendements. Quels sont ceux qui sont en cours. Qui sont contre, qui s'abstiennent, l'amendement est adopté.

C'est une demande de retrait parce que je partage l'intention simplement, ça vous a pas échappé je vois sénateur qui devait la majoration s'appliquerait à partir de 2022, et surtout se repérer.

Merci monsieur le président, alors là il s'agit je vous reconnais j'abuse un peu, mais d'un élargissement de l'assiette du crédit d'impôt, cinéma. Aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l'oeuvre et aux frais d'assurance destiné à couvrir les risques encourus à compter du 1er janvier 2021 pour permettent de renforcer l'efficacité. L'avis de la commission. ça va être une demande de retrait pour éviter les abus. Gouvernement. Je le retire. 2 amendements en discussion commune identique le 439 rectifié Madame Darcos. Alors là, il s'agit du crédit d'impôt cinématographique internationale enfin ce crédit d'impôt pour dépenses de production d'Oeuvres cinématographiques audiovisuelles concerne aussi les initiatives étrangères dont toute une partie de fabrication a lieu en France, il a prouvé son efficacité depuis sa création 2009 en attirant en France en 2019 un total de 245 millions d'euros de dépenses à la fois pour de grosses productions cinématographiques pour des séries TV et des Oeuvres d'animation autour de Studio et faisant appel aux talents français les projets internationaux sont d'une ampleur significative et nécessite une longue préparation, ainsi pour les films de 2022 à 2023, les décisions seront prises en 2021 donc, chers collègues, c'est un peu différent de ce qu'on a voté tout à l'heure, là on ne peut pas simplement le faire pour 2021 c'est une anticipation au moins même si, bien sûr, je ne veux pas que ce soit forcément pérenne mais que ça soit au moins jusqu'en 2023 et films d'animation ont en général une durée de production de 24 à 30 mois ils sont donc systématiquement à cheval sur au moins 3 années civiles les tournages de films sont anticipées au moins 18 mois à l'avance, en raison des castings et des préparations enfin les séries doivent être sécurisés sur plusieurs années, eu égard à leur réalisation sur plusieurs saisons, afin de pouvoir réutiliser les décors, équipements et figurants d'une saison sur l'autre la christianité économique a frappé de plein fouet l'ensemble de ces secteurs et en même temps si les tournages ont pu reprend progressivement en France comme dans certains pays, en fonction de l'amélioration de leur situation sanitaire les productions internationales sont cependant retardé notamment par l'incertitude pesant sur la réouverture massif des salles de cinéma des principaux marchés mondiaux, un grand nombre de projets ont déjà été décalés tant production sortir, repoussant d'autant les projets suivants dans ce contexte de décalage en cascade, les producteurs étrangers veillerons attentivement à leur capacité à supporter un glissement important de calendrier dans le pays choisi sans que celui-ci des conséquences trop importantes sur leur budget, notamment du point de vue fiscal rappelons que plusieurs pays propose à ses producteurs des avantages fiscaux attractifs, comme le Royaume-Uni, Canada, Allemagne sans limite dans le temps, le crédit d'impôt est bornée dans le temps et son extension ne peut porter que sur une période maximale de 4 ans, il a été prolongé par la loi de finances 2019 jusqu'au 31 décembre 2022 dans cette période d'incertitude que nous connaissons actuellement, il est indispensable de prolonger par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2024, faute de quoi les tournages qui seront mis en oeuvre en 2022 2023 seront décidées durant l'année 2021 échapperont à la France, telle est l'objet de ce prêt de cet amendement. 968 rectifié Monsieur non pardon Monsieur Oui, monsieur le président, cet amendement est identique au précédent, il a été très bien défendu par notre collègue Laure Darcos si vise à à repousser de 2 ans, le crédit d'impôt, qu'elle a évoqué précédemment. Avis de la commission Alors ce ce crédit d'impôt, comme ça a été évoqué par la sénatrice Laure Darcos est effectivement un élément clé de la relocalisation ces dernières années de la production cinématographique en France les éléments ont été donnés, je pense, donc évidemment on ait souscrit ce sera un avis de sagesse reste néanmoins que cette prolongation ne dépend pas uniquement de la volonté du législateur, vous le savez, on a besoin d'avoir l'avis de la Commission européenne, qui dans le passé, a remis en cause certaines évolutions de ce crédit appoint donc une prudence mais en ce qui me concerne c'est un avis de sagesse.

le dispositif est bien mais vu le contexte, il y a besoin d'un minimum d'anticipation et c'est une bagarre, des fois qui se joue à peu avec beaucoup de pays, on était dans une situation où même les tournages de films français, aller à l'étranger Belgique etc parce que c'était nettement plus économique, on a pris des mesures, ses revenus, et nous avons été avec cette mesure sur le cinéma étranger, nous avons en plus de localiser le cinéma français, nous avons attiré des grosses productions et des films étrangers, qui ont permis de de créer beaucoup d'activités, parce que quand il y a une machine lourde comme ça qui arrive dans une ville et c'est pas toujours pareil, ça. Pour beaucoup d'activité d'emploi mais aussi de de pour tous, pour le commerce caetera et ça s'est fait de façon importante, donc les effets visibles concret, on devrait faire ça plus souvent d'ailleurs pour dire si une mesure hé bien ou pas bien, c'est après l'avoir prise 2 ans après, c'est quoi le résultat bénéfice et coup hé bien là, c'était plutôt très positif, mais pour ça, continue, faut que cette visibilité sur 2 ans à cause de la crise, ce qui est proposé tout à fait responsable et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Je vais mettre aux voix, ces 2 amendements, quels sont ceux qui sont pour.

il consent généralement une avance minimum garanti versé aux producteurs et frais distribution sur des films à venir une fois le film achevé il en acquiert les droits, et assure l'édition, la promotion, la commercialisation de l'oeuvre, la distribution et donc un secteur d'activité à risque car les distributeurs engage des frais d'édition et de communication important pour des succès en salle très difficilement prévisibles, économie de prototypes dans un contexte sanitaire instable et des conditions d'exploitation contrainte lorsque les salles sont ouvertes juge d'accueil limitée distanciation physique, les perspectives de fréquentation du public sont plus qu'incertaines, compte tenu de l'investissement important que représente la sortie d'un film, cette incertitude peut amener les distributeurs à retenir des films dans l'attente des perspectives meilleures or une offre large régulière de films dans les salles, y compris de films populaires étrangers sera nécessaire à la reprise de l'activité, ça la fréquentation à la sortie du confinement contenu du contexte de la crise des mutations de fonds sont à l'oeuvre avec le constat d'un effondrement sur le marché secondaire des distributeurs en VOD vidéo physique diffusion TV sans que les ventes aux plateformes et pris encore le relais, le développement du piratage pèse également très lourd, il se développe particulièrement dans les périodes de confinement, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs, l'Hadopi nous l'a confirmé dans ce contexte, et en attendant que le marché trouve de nouveaux équilibres, l'État a vocation à intervenir pour rendre l'équation économique distributeurs plus soutenable et les inciter à commercialiser des films de façon régulière tout au long de l'année 2021, permettant ainsi d'approvisionner régulièrement les salles de cinéma en contenu, c'est un enjeu culturel majeur, ainsi qu'un soutien nécessaire à toute la diversité des films ce crédit d'impôt prévues par le présent amendement sur les frais de sortie des films générera des retombées positives pour l'ensemble des fournisseurs qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures, concepteur de bandes annonce attaché de presse agence de communication tout un tissu d'entreprises directement touchées par la crise pour les médias, dont les ressources pour publicitaires ont été affectées par la crise pour les salles de cinéma qui dépendent des distributeurs pour la programmation pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé distributeurs pour financer de nouvelles Oeuvres en avec des montants garantis. comment dirais-je, ce projet de loi de finances répond, me semble-t-il, l'absence de dépenses fiscales dédiée avec l'élargissement du Champ d'intervention des Sofica qui est prévue à l'article 42 elle je précise en plus qu'à ce nouveau dispositif fiscal s'ajoutent les montants prévus par le plan de relance plus 17 millions d'euros qui devrait donc ainsi être dédié à la relance de l'exploitation en salles, raison pour laquelle, selon moi, via des aides à la distribution, selon moi, l'amendement est satisfait, d'où la demande de retrait. Madame Darcos. une incertitude sur le chemin, le plan de relance pour le CNC, qui devait en effet de la TSA les exploitations puisque, en fait, à l'Assemblée nationale a été votée, je ne m'en reparler tout à l'heure, un amendement qui exonéré la TSA les les exploitants de salles jusqu'à la fin de l'année, ce qui est un manque à gagner de près de 20 millions d'euros pour le CNC, donc du coup, le CNC ne pourra pas contribuer, en tout cas à ce à à cet effort-là dans le plan de relance actuellement, telles que le texte est voté au PLF 2021. Vous le maintenez, monsieur Assouline. et qu'on trouve une mesure plus juste et plus plus cohérente qui aurait d'ailleurs coûter moins cher en même temps, bon, de toute façon quand ça vient au CNC, cette taxe elle repart vers les salles. Mais c'est une question de trésorerie qui va avoir la trésorerie quand ça vient d'abord au CNC, le trésorier le le CNC, la trésorerie si ça vient directement vers les salles de la et en ce moment tout le monde a des problèmes de trésorerie alors. Le CNC nous dit il faut faire ça. Et puis les salles nous disent : ben non, non, non, non, non, ne faites pas ça. Moi ce que je pense c'est que nous, on doit être dans quelque chose qui ait du sens. On a exonéré de taxe parce qu'il y avait une situation où on n'avait plus le droit d'aller au cinéma, donc les salles étaient complètement asphyxiés donc on peut considérer que cette exonération a lieu sur les mois de confinement, pas sur l'ensemble de l'année. et donc ça coupe la poire en deux hein, si on fait comme ça, c'est-à-dire que, il y a une partie qui vient au CNC directement ça allégera leurs problèmes de trésorerie peut-être et puis une autre partie qui vient directement au sol qui ont été dans une extrême difficulté qui ont besoin d'aide, mais au final, de toute façon. Il faut savoir que cette taxe quand elle est prélevée par le CNC, elle va en partie au sol de, de, de, de, de, de participation des salles, elle revient vers elle, donc je ne sais pas si j'étais Claire, je pense que oui, pour ceux qui m'ont suivi, mais en tous les cas, peut-être que je ne sais pas s'il y a encore des possibilités de navettes de de discussion en CMP, ailleurs on peut trouver une mesure juste exonération pendant les mois de confinement, ce qui couperait la poire en 2, de ce qui est aujourd'hui envisagée. Je me trouverai cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Il n'est pas adopté.

Un amendement en 63 monsieur Beuchere. Monsieur le président, Monsieur le Ministre je ce rapporteur général, mes chers collègues, c'est un amendement frappé du triple saut du bon sens, de la cohérence et que la gratuité et au surplus du renfort du pouvoir de contrôle du Parlement, il va donc être adopté à l'unanimité, il s'agit, en termes de parallélisme des formes pour le nouveau crédit d'impôt sur la musique liés dans l'eau à la création du Centre national de la musique que soient publiés les agréments à la, à l'image de ce qui se fait pour le CNC c'est donc juste le le CNM, qui doit publier les agréments. C'est un avis favorable. Des femmes défavorable car contrairement secret fiscal. Je vais mettre aux voix l'amendement, il n'y a pas d'explication de vote, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent il est adopté. 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 249 Madame Dumas.

Merci monsieur le président, il s'agit de de créer un un crédit d'impôt en faveur de l'édition musicale, les éditeurs musicaux sont un partenaire évidemment essentiel dans le monde de la musique, moins connu que les auteurs compositeurs ou que les producteurs, mais pour autant, les auteurs ont besoin du secteur de l'édition musicale, qui joue un rôle très important dans l'accompagnement des artistes et des Oeuvres, il souffre beaucoup de la crise liée au Covid ils était déjà d'ailleurs fragilisée et c'est pourquoi cet amendement près prévoit de de les soutenir via un mécanisme de crédit d'impôt. Avis de la commission. une demande de retrait au profit des amendements suivants le 84 627 747260 qui sont en discussion commune et convergents. Donc 3 amendements identiques le 84 le 627 le 744 le 1260 le présent amendement propose donc la mise en place d'un crédit d'impôt en faveur de l'édition musicale visant à soutenir la création d'Oeuvres musicales et le développement de carrière d'auteurs de compositeurs d'Oeuvres musicales par les éditeurs de musique dans ce secteur, l'éditeur étant en tant que partenaire de l'auteur-compositeur, le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l'exploitation permanent du suivi d'une oeuvre les renvois explicite du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession, témoigne du caractère protéiforme et fondamentale du rôle de l'éditeur musical en développant les Oeuvres la carrière de leurs auteurs compositeurs, l'éditeur soutient également la création des Oeuvres musicales et mutations du marché de la musique ont entraîné une réduction sensible des moyens d'action, les entreprises d'édition musicale et l'équilibre financier déjà fragile de ces dernières a été dégradé par la crise sanitaire et économique, l'érosion de la capacité de financement des éditeurs s'est traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard aux risques plus importants représentée par les projets avec les nouveaux talents, le crédit d'impôt participerait donc à la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents, il accompagnerait l'activité des sociétés d'édition musicale à leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière et c'est d'autant plus que l'on va l'engagement de l'éditeur se situent souvent en amont des projets dans un 1er cycle de développement pendant lequel le risque est maximal il permettrait également de rendre les sociétés d'édition musicale plus compétitive au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de langue française, le tout en bénéficiant aux finances de l'État plusieurs critères au Canada encadre concentre le Champ d'application du présent projet le crédit d'impôt basé sur le contrat de préférence, il ne concerne que les auteurs nouveaux talents tient compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles notamment soutien la création et au développement de carrière égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées, aussi, de contrats de préférence éditorial agréés, il s'applique : d'une part aux sommes versées jusqu'au 31 décembre 2024, dans la limite d'un plafond de crédit d'impôt de 500000 euros par entreprise et par exercice et, d'autre part aux dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021. Monsieur George, pas pour le 627. C'est le même, il a été très bien présentés, voilà, on insiste sur ce milieu de l'édition musicale qui ne doit pas être l'angle mort du monde de la musique, on connaît plus d'autre bout de la chaîne que que ce que le monde des éditeurs phonographiques.

Oui je je présente s'il s'agit du même amendement mais Madame Sylvie Robert, qui a proposé cet amendement de mon groupe se bat, particulièrement pour cette filière et tenait à ce que cet amendement soit porté devant l'hémicycle, je ne vais pas dire et répéter ce qu'à ce qui a déjà été très bien exposé au mot près, on va dire

disons à la sensibilisation de, de, de, de l'attention qu'on doit porter au monde de la musique en général il y a eu un, un appel à l'aide du président de la Sacem, ces dernières heures, qui explique que la situation est dramatique, il dit : ce qui nous font rêver, vont-ils continuer à vivre parce que on en est là, c'est pas quelque chose, disons d'extrapoler d'exagérer c'est concrètement la possibilité, si on ne soutient pas par tous les bouts d'ailleurs cette filière mais ce bout de l'amendement est est tabou important et est souvent un angle mort, comme l'a dit, Julien Bargeton, hé bien on va voir les conséquences dans les années qui viennent, en terme de, de qualité des productions, terme de diversité parce que c'est souvent dans ce cas-là, les petits qui meurent et donc cet amendement va dans le bon sens et il est identique aux autres. Avis de la commission. Alors je l'ai dit, en rendant la vie tout à l'heure je vais éviter de rallonger les débats, c'est un avis de sagesse pour l'ensemble de ces amendements. Le gouvernement. Je vais mettre aux voix, ces amendements identiques, quels sont ceux qui sont pour. Contre qui s'abstiennent, ils sont adoptés. 3 amendements identiques. Madame Darcos pour le 80 rectifié. Merci monsieur le président, alors celui-ci pose le principe général, une possibilité d'exonération de cotisation foncière des entreprises pour les très petites entreprises de musique enregistrée et d'édition musicale dans les communes volontaires, l'article 1464 M du code général des impôts prévoit déjà cette exonération pour les disquaires indépendants qui favorise à l'accès à la culture sur l'ensemble du territoire une extension aux petits producteurs phonographiques et éditeurs de musique, dans le contexte de la reprise post-Covid contribuerait à soutenir la création de la diversité musicale au cours des 3 étapes se sont que sont l'exploitation de leur son enregistrement et sa distribution, ces entreprises déjà fragilisées par la crise continueront d'en subir les conséquences de manière différée, l'année prochaine lors de la répartition des droits d'auteur et des droits voisins au Tir de l'année 2020, de fait, en raison de la fermeture des lieux publics et de l'effondrement des ventes de supports sur lesquels sont majoritairement assise la rémunération équitable et la la copie privée, l'année 2021 s'annonce très difficile pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent, cela se traduira à moyen terme, à la fois par une baisse de revenus structurant par une attribution des aides à la création une attrition pardon des aides à la création, servi par les organismes de gestion collective dans un contexte marqué par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 septembre 2020, qui divise par 2 les sommes mobilisables à cet effet, moins 25 millions d'euros par an dans ses perspectives, la mesure d'exonération proposée aura pour effet, dans les communes volontaires de baisser les charges fiscales locales, des entreprises les plus fragiles du secteur et surtout de favoriser le maintien et le développement de la vie culturelle dans ces territoires. Monsieur Bargeton. Oui, merci Monsieur le Président, c'est le même pour un indique ainsi, c'est sur le fait que il s'agit des des très petites entreprises et donc il s'agit bien là de défendre vraiment la diversité puisque dans ce monde de de de l'édition phonographique-là on se focalise sur les TPE et donc sur ce cet écosystème qui permet de faire vivre une diversité d'auteur-compositeur. de un avis de sagesse dans la mesure où l'exonération être évidemment facultatives donc on laisse aux collectivités la possibilité, la faculté d'accorder ces exonérations. Je vais mettre aux voix, quels sont ceux qui sont pour. Qui sont contres qui s'abstiennent qui sont adoptés. à l'article 43 obtiennent un amendement en France présenté par monsieur le rapporteur. est un amendement pardon qui propose de supprimer l'article en ce qu'il propose finalement de rétablir une réduction d'impôt pour les autres entreprises de presse à la fois les exploitants, les éditeurs pour tout vous dire, monsieur, je pense que le l'amendement êtes et est mal rédigé et je pense qu'il est également inapproprié en ce qu'il vient à distinguer les exploitants des éditeurs et même si c'est une dépense fiscale qui n'est pas très importante, on l'a vu souvent inférieur à un 1000000 d'euros, le fait de vouloir à ce stade, rétablir ainsi cette dépense fiscale ne me paraît pas justifié, raison pour laquelle je propose la suppression de l'article. Merci monsieur le président, le gouvernement et est défavorable à la suppression de l'article, dans la mesure où nous avons soutenu son intégration lors de l'examen à l'Assemblée nationale, vous avez évoqué un certain nombre de points, nous avons aussi évoqué en aparté, donc d'ici là, navette, nous, nous regarderons comment veiller à ce que ces articles soient parfaitement opérationnel par rapport à l'objectif que nous avons mais défavorable à la suppression. Je mets aux voix cet amendement, quels sont ceux qui sont pour. Le sens qui sont contres qui s'abstiennent. L'amendement est adopté et l'article 43 et c'est au c'est supprimé. Un amendement 277 rectifié Madame Marcos. Merci monsieur le président, le présent amendement vise à instituer un crédit d'impôt au bénéfice des particuliers qui acquièrent des Oeuvres d'artistes vivants des arts visuels, il permet de compléter les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire qui, bien que nécessaires répondent de manière partielle aux difficultés qu'il rencontre en raison de la fermeture de tous les espaces de vente et de diffusion, l'annulation d'événements ou encore l'intervention d'accueil du public dans les ateliers, cet amendement tend à encourager la création contemporaine en matière d'arts visuels graphiques et plastiques à soutenir le marché de l'art et promouvoir la démocratisation culturelle de l'art contemporain. Avis de la commission. le dispositif oblige par ailleurs les entreprises à exposer l'oeuvre au public, ce qui n'est par contre pas retenu dans la rédaction de votre amendement et c'est une demande de retrait. Madame Marcos pour le 986 sièges. Je vous promets qu'après on passera à autre chose, mais avoir une demi-heure sur la culture sur l'ensemble du PLF, je pense que c'est, c'est finalement voilà assez, oui mais bon en partie. Le présent amendement a pour objet d'améliorer la fiscalité des librairies, vous savez, ça me tient particulièrement à coeur et des propriétaires de locaux commerciaux loués à des libraires pour ces derniers, il est proposé une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition expresse qu'ils s'engagent à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyers applicables lors de la prise d'effet du bail à renouveler, y compris si celui-ci a une durée supérieure à 9 ans ainsi que lors de chaque révision du loyer triennal, considérant que le loyer représente l'un des postes de dépenses plus élevé de lors de 5 à 10 % du chiffre d'affaires menaçant à court terme, l'existence même d'une offre culturelle de qualité en centre-ville, une telle mesure devrait être de nature à stabiliser la charge pesant sur les libraires, il est également proposé une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises au bénéfice des librairies disposant du Label lire afin que les librairies labellisées librairies de référence libre et non labellisés relevant de la catégorie des petites moyennes entreprises puissent également bénéficier d'un soutien des collectivités territoriales, il est donc proposé que ces dernières, la faculté de les exonérer à titre facultatif sur délibération de portée générale, chute de vous dire. Que l'émoi qu'a suscité la fermeture des librairies ou la non-réouverture des librairies, fait que c'est des sujets qui me tiennent à coeur, même si je sais, j'entends déjà des membres de la commission des finances, dire que c'est abusé mais c'est symboliquement très important pour nos libraires. Avis de la commission. Les difficultés rencontrées par le secteur de confinement chute dramatique du chiffre d'affaires, évidemment il faut réfléchir, essayer de trouver des dispositifs innovants, puisque finalement si on peut aider ces entreprises à traverser le la crise, pourquoi pas, mais dans la 2ème partie de l'amendement, vous visez l'exonération de cotisation foncière des entreprises, là c'est plus complexe, une exonération facultative est déjà prévue pour les librairies indépendantes dites de référence votre amendement propose une extension de cette exonération facultative aux librairies labellisées librairies de référence et aux librairies non labellisés relevant de la catégorie des PME, là encore, cela je le dis, relève du libre choix des collectivités cette extension en fait, elle est en plus ce n'est pas totalement symétrique parce que l'exonération des librairies indépendantes de référence deviendrait dans le même temps, obligatoires, ce qui induit, et vous le savez, une fois que c'est obligatoire, une baisse de ressources pour les collectivités, sans aucune compensation demande de retrait.

Il n'est pas adopté. Je mets aux voix, l'article 43 perd des sièges, quels sont ceux qui sont pour.

à l'article 43 DCS je de amendement de rédaction globale qui font l'objet d'une discussion commune le 11 31, monsieur le rapporteur.

cet amendement prévoit le renforcement et le prolongement du crédit d'impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique, en effet, cet outil est essentielle pour accompagner la transition de l'agriculture vers des modes de production qui soient vertueux, l'agriculture biologique est un outil de la transition agroécologique reconnue depuis longtemps et comme l'a rappelé le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l'agro- écologie qui affirme l'efficacité de l'agriculture biologique définie définie comme je cite la plus performante d'un point de vue tant économique qu'environnemental, aujourd'hui, l'agriculture biologique est aussi un mode de production, identifié par les consommateurs, pour lesquels la demande augmente fortement, aujourd'hui encore, nous importons une part beaucoup trop importante de notre alimentation bio, faute de soutien à son développement en France, dans le même esprit que l'aide au maintien, ce crédit d'impôt se justifie largement par les nombreuses externalités positives associées à l'agriculture biologique, tant sur la qualité de l'eau que celle de l'air, la protection des pollinisateurs la préservation des sols, la réduction de la la qualité la qualité de l'alimentation, la santé humaine de plus alors que le présent projet de loi prévoit un crédit d'impôt de 2500 euros pour les exploitations certifiées haute valeur environnementale, il est cohérent de revaloriser le crédit d'impôt bio dont le cahier des charges est bien plus exigeants en terme environnemental, la haute valeur environnementale, nous en discuterons à l'article suivant n'a rien à voir avec les exigences du bio, il faut véritablement maintenir un différentiel dans le crédit d'impôt pour garder une une distinction claire entre ces 2 certifications et de renforcer le soutien à l'agriculture biologique en portant à 4500 euros le crédit d'impôt bio, enfin, cet amendement propose de sécuriser ce crédit d'impôt en le prolongeant jusqu'en 2024 en effet, alors que le plan Ambition bio fixe un objectif de 15 % de la surface agricole utile conduite à en agriculture biologique en 2022 que le Pacte Vert pour l'Europe fixe pour 2030 25 % des Terres en bio, il est important de donner un cap et une visibilité en prolongeant pour 4 ans, le crédit d'impôt bio à l'heure où tous les 2 ans, des inquiétudes planent sur son renouvellement.

mais vous avez donné un avis défavorable je le rappelle, un amendement de crédits permettant de réintroduire des aides au maintien pour les exploitants agricoles en bio aide que le ministère de l'Agriculture a décidé de ne plus attribuer, par exemple, au contraire des agences de l'eau et de partenaires européens, dans le cas du plan de relance le bon niveau du crédit d'impôt bio est toutefois, me semble-t-il difficile à déterminer, elle est prochain règlement financier de la PAC à venir ne sont pas encore adoptée et je pense enfin qu'il vaut mieux borner la prolongation du crédit d'impôt à 2022, pour des raisons qu'on a déjà évoqué au long de nos précédents précédents travaux un avis défavorable. Ministre. L'avis est défavorable sur l'amendement de monsieur l'abbé pour les raisons évoquées par monsieur le rapporteur, j'ai donné tout à l'heure, un avis de sagesse sur l'amendement de monsieur le rapporteur, que j'avais un doute sur une question de rédaction en réalité il est favorable.

attendu qu'elle a fait ses preuves et qu'on a des engagements nationaux qui ont été prises sur sur 2022, on est loin du compte, alors on voit arriver, moi je ne veux pas lancer le débat là-dessus, mais, mais quand même, on voit arriver la montée en puissance de l'de l'agriculture à haute valeur environnementale, ce n'est pas le même niveau, ce n'est même pas une étape pour l'évolution vers l'agriculture bio et quand on dit des ambitions bio, ce sont des ambitions bio et pas l'ambition européenne et bio également et pas achevée mais on voit doucement glisser un mouvement comme ça pour faire en sorte que le Label environnemental agro- equal écologique soit simplement la HVE et je tiens à dire que cette absolument inacceptable pour le climat pour la biodiversité pour les équilibres environnementaux et aussi pour les agriculteurs parce qu'que elle, elle envisage le développement industriel de l'agriculture et pas l'agriculture paysanne que nous demandons de nos voeux.

Cet amendement vise à supprimer le crédit d'impôt pour les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale introduit sans étude d'impact, par voie d'amendements à l'Assemblée nationale en effet cette certification n'a pas fait ses preuves, puisque les retours terrain montre que de nombreuses exploitations agricoles obtiennent la certification HVE sans véritablement améliorer leurs pratiques en exploitant les failles du cahier des charges, telle qu'il est actuellement rédigé à titre d'exemple sur la question des finaux des phytosanitaires, la haute valeur environnementale n'empêche pas l'utilisation de produits qui sont classées cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, de même la certification peut être obtenu par le calcul d'un ratio de 30 % entre le chiffre d'affaires et le montant des sommes allouées à l'achat des pesticides ainsi les exploitations qui ont des chiffres d'affaires importants peuvent bénéficier de la certification sans changer du tout leur pratique en clair, celui qui, il y a plus d'argent peut utiliser plus de pesticides, et on trouve ainsi, sans surprise, que 80 % des fermes HVE sont des exploitations viticoles, c'est logique, imaginons ce que représente 30 % du chiffre d'affaires d'une exploitation de Cognac en termes d'achats de pesticides l'élevage le cahier des charges HVE ne comporte aucun élément sur des pratiques clé permettant d'engager réellement les fermes dans la transition agro-écologique par exemple il ne comporte rien sur les prairies et leur gestion sur l'accès à l'extérieur des animaux ou encore le pâturage, il n'y a aucun critère sur le bien-être animal, notamment sur la densité dans les bâtiments, ni aucun élément sur la provenance ou la qualité de l'alimentation des animaux ou encore sur la réduction des antibiotiques qui sont pourtant des enjeux stratégiques pour la pour la transition des élevages, le cahier des charges HVE et par ailleurs, complexe et peu lisible, il peut être intéressant de valoriser et d'encourager, évidemment, des pratiques intermédiaire entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, ce qui est l'objectif affiché de la VE mais son cahier des charges n'est pas à la hauteur d'une étape intermédiaire.

pour décortiquer et finalement dire toutes les insuffisances, voire le mal que vous pensiez de ce qui est des charges, moi je pense qu'il faut regarder plutôt le verre à moitié plein, c'est-à-dire se dire que ça démontre bien, en tous les cas qu'il y a une volonté, une aspiration avec des étapes se mettent progressivement en place pour faire gagner la conscience écologique à tous les secteurs d'activité, y compris, à commencer par l'agriculture, qui d'ailleurs n'a pas attendu non plus, ce crédit d'impôt, mais c'est un un 1er pas donc un avis défavorable.

Oui, vous comprendrez que j'insiste. Et j'insisterai plus que jamais cet amendement, cet amendement vise à encadrer le crédit d'impôt type de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale instaurée par l'article 43 du duo des siestes introduit par voie d'amendements à l'Assemblée nationale, sans étude d'impact, il vise à amorcer en lien avec la création de ce crédit d'impôt, une réforme du cahier des charges de la haute valeur environnementale qui n'offrent aujourd'hui pas de réelle garantie d'évolution vers des pratiques vertueuses sur le plan de la transition agro-écologique. Si la HVE devait être soutenue financièrement par les politiques publiques, il conviendrait alors de faire évoluer fortement et rapidement son cahier des charges vers une meilleure prise en compte de l'environnement et du bien-être animal, ce cahier des charges devraient également pour les auteurs de cet amendement inclure des critères sociaux, notamment sur le partage de la valeur puisque la modification de leurs pratiques par les agriculteurs ne peut se faire sans équité économique : le crédit d'impôt serait ainsi prévue pour 2022 pour permettre une évolution du cahier des charges en 2021 pour les mêmes motifs de faiblesse de cahier des charges. Cet amendement considère que le crédit d'impôt proposé par le présent projet de loi est trop élevé, en effet, le crédit d'impôt, il y a cette certification et de 2500 euros contre seulement 3500 euros pour le crédit d'impôt bio alors que le cahier des charges et bien plus exigeants en forme, nous jugeons que l'art et autres trop activités de ce crédit d'impôt qui a proposé à toutes les exploitations certifiées depuis 2011 et problématique, ce dispositif est supposé d'après l'exposé des motifs de l'amendement atténuer le coût administratif de cette certification environnementale et encouragé à la transition agroécologique quittait le cas pourquoi ils rendent éligible des exploitations qui ont déjà franchi le pas vers cette certification, les députés, auteur de l'amendement évoque pour justifier cette rétroactivité la crise il y a l'épidémie Covid 19 ceci, interroge, nous interroge sur la certification HVE HVO qui ne présentent pas de lien avec les difficultés économiques qui seraient liés à la situation sanitaire. Ou se 45 Madame Carrère. Merci monsieur le président, la France a décidé d'accélérer la transition écologique de son agriculture, nous avons en particulier des engagements à travers la PAC qui dit de plus en plus les aides aux efforts de préservation de l'environnement, les agriculteurs sont ainsi placés devant un défi produire mieux, tout en restant compétitif dans ces conditions, la mutation agro-écologique implique de nouveaux investissements, bien souvent, une hausse des coûts de production parfois un ralentissement de la production et presque toujours les démarches administratives supplémentaires dans la période de crise sanitaire et économique que nous traversons, ces contraintes deviennent difficiles à tenir, la création d'un dispositif fiscal HVE s'inscrit dans la politique d'accompagnement de la conversion à l'agroécologie, je rappelle que le gouvernement a fixé un objectif de 15000 exploitations certifiées HVE à la fin 2000 22 et de 50000 en 2030, cependant, avec un crédit d'impôt HVE limitée à 2500 euros, on crée un déséquilibre avec le crédit d'impôt pour les exploitations converties au bio dans dans le montant est passé à 3500 euros depuis la loi de finances pour 2018 pour une plus grande équité fiscale et nous proposons par cet amendement de fixer le dispositif fiscal HVE également à 3500 euros. Merci si on. Avis de la commission, c'est ni plus ni mois que ce qui est proposé par le gouvernement, donc 2 avis défavorables laissons honnêtement, déjà, les choses se mettre en place, il sera temps après, parce que si chacun y va de son chiffre pourquoi pas 5 1000, 10 1000, et pourquoi pas rien du tout.

Oui, beaucoup de nos agriculteurs, quel qu'il soit, quels que soient leur pratique se retrouvent en difficulté avec ce modèle. Donc, cet amendement, qui devrait faire consensus, cette fois, vise à faciliter la prise de congé des agriculteurs en augmentant le montant du crédit d'impôt permettant de financer le recours aux services de remplacement, j'avais proposé cet amendement partie hein du PLF, il avait été jugé intéressant mais allant trop loin au niveau de la prise en charge prévu je propose donc cet amendement remodelé et moins ambitieux mais qui sera néanmoins très utile pour permettre aux agricultrices et agriculteurs de partir en vacances, pour rappel, actuellement ce crédit d'impôt permet aux éleveurs et aux paysans, contraint à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d'un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congés dans la limite de 14 jours par an, cet amendement propose de passer ce taux de financement à 75 pour la première semaine de congé puis de rester à 50 % en ce qui concerne la 2ème semaine en effet encore trop d'agriculteurs ne prennent aucun coup aucun congé sur la niche et même la majorité du fait de contraintes économiques, cette mesure aura plusieurs effets positifs, elle permettra de renforcer la l'attractivité du métier d'agriculteur dans un contexte où l'agriculture française est confrontée à l'enjeu crucial du renouvellement de générations, alors que le nombre d'exploitations, baisse de 1 à 3 % par par an, il nous faut redonner l'attractivité à la profession, le métier d'éleveur est particulièrement concernée avec un vieillissement de la population, une surcharge de travail, générant fatigue physique et épuisement psychologique, ainsi qu'un rapport différent des nouvelles générations aux contraintes de l'astreinte de plus cet amendement permettra de créer de l'emploi stable et sécurisée bénéfique pour la dynamique des territoires ruraux, selon le service de remplacement, la mise en place de crédit d'impôt a permis déjà de développer fortement l'accès au congé les remplacement pour congés, passant de 80000 journées à 180000 journées, ce crédit d'impôt serait donc à Louviers efficace à la création d'emplois, il est également il que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes avec cette mesure, les salariés concernés resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent et se ruent, ce l'or l'opportunité d'installation et sera bénéfique pour le le renouvellement des générations, je vous remercie. Monsieur le sénateur, la ce sera une demande de retrait, vous avez bah oui, parce qu'à un moment donné, pour une fois, je le dis, moi je le fils et frère de l'agriculteur qui s'exprime devant vous, mais comme d'autres, je pense qu'il faut garder en terme de crédits d'impôt dès une proportionnalité et 50 % de crédits d'impôts, ça me paraît déjà un bon niveau, surtout pour des services et de 10 de remplacement, je rappelle également que nous avions évoqué, je crois que c'est un des sujets sur lesquels il faut travailler, c'est plutôt également la durée pendant laquelle les agriculteurs peuvent ou pourraient partir parce que quand vous avez je je partage une bonne partie des éléments d'appréciation sur la difficulté du métier aujourd'hui notamment d'éleveurs mais je pense aussi que dans les solutions sur lesquelles il faut travailler et qui ne dépendent pas malheureusement que la France, c'est que nos paysans puissent retrouver des revenus décents c'est ça le combat qu'il doit être le nôtre, il passe par un ensemble de réflexions mais je, je vous demande le retrait pour l'amendement, revue et corrigée par rapport à celui la version vous aviez déposé dans le PLF. Défavorable, malgré les ajustements apportés par monsieur le sénateur. Monsieur l'abbé. Non seulement je ne suis pas satisfait par la demande de retrait, mais je suis un peu outré,

sur la et on a, on a travaillé les uns et les autres sur la question de la détresse du monde agricole avec avec Henri Cabanel notamment, c'est la solitude, le manque d'ouverture, le manque de, de, de, de décompression fait que beaucoup se retrouvent avec les avec les dettes avec tous ces aspects-là, alors la question de dire oui, bah, il faudrait que les que les agriculteurs un un revenu décent et à ce moment-là il pourrait prendre des vacances, mais ça c'est un peu un voeu pieux, rien n'est fait pour cela, la loi Egalim est un échec total au niveau de, au niveau du revenu des agriculteurs, il importe de le dire, mais il y a ceux qui souhaitent sans le dire qu'il y en ait encore moins pour que les fermes soient encore plus concentré et c'est pas notre point de vue, c'est pour ça qu'on défend avec force merci. merci. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues, je vais défendre moi cet amendement parce que je trouve effectivement que le problème posé par Joël Labbé est une vraie difficulté aujourd'hui dans nos zones rurales, le monde agricole fait face à à à la détresse, parce que les prix ne sont pas suffisamment rémunérateur et on sait bien tous ceux qui vivent à la campagne, combien le métier est difficile et prenant combien il est engageant un c'est un travail pour les éleveurs laitiers par exemple, 7 jours sur 7, et il est absolument indispensable que ces producteurs que ces agriculteurs puissent prendre des congés ce qu'ils ne font pas tous y compris pour des et en particulier pour des raisons financières, compte tenu du du niveau de rémunération issus des des productions, le prix du lait par exemple c'est 34 centimes le lait, le litre, inutile de dire qu'ils ne gagnent pas leur croûte avec ça, c'est pas possible, donc il faut trouver des systèmes qui permettent d'assister à ce que les agriculteurs puissent, comme tous les autres effectivement prendre des des congés donc, même si le système, il peut paraître, je dirais, élevé en termes de crédits d'impôts mais 75 % pour la forme de d'abonnements pour la première semaine, je trouve que c'est pas mal, si ça peut avoir ce caractère incitatif qui permettra effectivement aux agriculteurs de pouvoir comme toute tous les concitoyens de pouvoir bénéficier de congés.

alors même si la loi Egalim elle n'est pas parfaite, il faut sûrement travailler pour que, qu'elle s'améliore, mais, mais les agriculteurs ne ne demande pas l'aumône cas que je connaisse et demande pas à ce qu'on leur prenne en charge leurs vacances, ils ne demande pas à ce que l'on l'envoie dans des comités d'entreprise ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui ment, il demande à ce qu'on trouve les solutions pour leur donner des perspectives sur l'avenir et qu'ils gagnent leur vie, alors donc je suis contre cet amendement, vous l'avez bien compris. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc je viens en soutien pour dire que nous allons voter cet amendement oui certes les et et c'est absolument indispensable que les agriculteurs puissent vivre de leur de leur activité, mais il y a urgence, on le sait, puisque les agriculteurs ne ne prennent pas la plupart d'entre eux de congés et s'il souffre donc psychiquement aussi de leur situation, donc je me moi il me semble que c'est une bonne mesure pour pallier un temps les problèmes qui devront être étudiée plus profondément, plus finement par la suite, je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'amendement, elles sont ceux qui sont pour.

n'est pas adopté. Je mets aux voix, l'article 43 perd des sièges, quels sont ceux qui sont pour. Qui sont contres qui s'abstiennent, l'article est adopté.

Oui, merci, alors je me suis intéressé à cet article parce que j'ai trouvé que le le dispositif avait un petit peu gadget quant aux regardez c'est-à-dire que venir diminuer la prime d'assurance quand on achète un véhicule électrique et l'idée derrière, j'ai bien compris que c'était d'inciter à l'achat de véhicules électriques, il me semble qu'il y a quand même un gros décalage entre la petite incitation qu'on donne sur la prime d'assurance et le surcoût d'achat d'un telle véhicules donc déjà ma première remarque et de dire que ce dispositif ne viendra aider que ceux qui peuvent déjà acheter un véhicule électrique, donc vraiment déjà les ménages les plus aisés, ensuite j'ai quand même un 2ème problème qui est que la prime d'assurance, son coût est notamment en fonction de la qualité du conducteur, donc venir cacher le signal prix en venant diminuer, enfin sauf à ce que vous m'amenez des statistiques qui montrent qu'un conducteur de véhicule électrique et bien meilleur conducteur qu'un véhicule de type diésel ou thermique, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'objets et, enfin, j'ai été regarder l'exposé des motifs pour voir si les auteurs de l'amendement était venu dire ce qui allait se passer pour sa diminution cette diminution, pardon de taxe supplémentaire : ben non, ils ne le disent pas, et donc la conséquence va être une diminution des financements qui sont apportées au départements pour le financement des services départementaux d'incendie et de secours à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les contrats d'assurance-maladie ainsi qu'au Conseil national des barreaux pour les contrats de protection juridique, donc j'ai un peu le sentiment Monsieur qui va peut-être arriver ce qui est arrivé avec l'article 2 du PLFR numéro 4, à savoir que sur un argument de maintenir les recettes de la fuite, on est venu des diminuer les recettes des collectivités donc pour toutes ces raisons, il me semble sage, de supprimer l'article 43 4 quater des siècles.

Mais ce dispositif, il constitue aussi et quand même une aide à l'achat d'un véhicule électrique, je pense qu'il faut effectivement faire attention aux effets d'affichage parce que, aujourd'hui, il y a pas d'abord de lien de corrélation étroite entre l'ambition écologique et l'aléa qui fait que les tarifs d'assurance sont fixés pour l'assurance automobile en fonction de la réalité des risques et des zones de circulation et non pas il y a pas par exemple d'assurance alors la le propose pour l'électrique ça oublie l'hydrogène ça oublier un certain nombre de mode de carburation plus propres, ce qui est dommage et il y a donc aucun lien en fait entre la réalisation du risque et puis cette réduction et puis peut-être aussi je je voudrais insister sur le danger de ces mesures est-ce que finalement elles vont être temporel et surtout temporaire. Et évidemment, le réveil pourrait être douloureux quand il faudra revenir à la fin de du dispositif de finalement de de réduction du montant de la prime, enfin, je veux vous faire part de de l'État un peu du marché, le, le prix moyen d'achat d'un véhicule électrique neuf comme la Zoé était d'environ 20000 euros. Aujourd'hui la moitié des propriétaires sont âgés de plus de 55 ans et vivent très majoritairement en zone urbaine, je dis ça parce que j'entends aussi la volonté affichée est pas caché d'ailleurs de dire il faut apporter des des réponses à la mobilité et des réponses évidemment propres mais ça veut aussi dire aujourd'hui que, faute d'avoir suffisamment d'équipements présents sur la totalité des territoires, ce dispositif risque au moins dans un 1er temps de taper complètement à côté de la cible. Il est défavorable, comme l'a dit Madame la sénatrice, c'est une incitation, parmi d'autres à l'achat de véhicules électriques qui vient s'ajouter aux primes que le gouvernement a mis en place pour la conversion. Explications de vote je met aux voix l'amendement, quels sont ceux qui sont pour.

Quels sont ceux qui sont contre. Qui s'abstiennent, l'amendement est adopté et l'article 43, peur des est supprimé. Monsieur le Ministre, vous voulez paroles. Un un mot pour prendre acte du résultat, c'est une mesure qui était proposé par la Convention citoyenne ce expliquait que le gouvernement l'avait intégré. gouvernement l'avait intégré. Monsieur le ministre, vous avez la chance d'avoir ici un peu moins que 150 citoyens mais ce sont des sénateurs citoyen également et vous le savez. Un amendement 14 82 présenté par monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a une espèce de convergence des temps et non pas des luttes puisqu'au moment où je présente cet amendement qui vise à conforter la position du Sénat à l'endroit des.

aujourd'hui il y a une absence en tous les cas où une défaillance du secteur des assurances parce que ce sont la plupart du temps des risques non couvert les questions de de la question, et notamment le risque de pandémie, mais pas seulement nous avons mis en place et votée au mois de juin, le 2 juin une proposition de loi à l'unanimité des suffrages exprimés avec quelques principes simples: apporter un dispositif par lequel nous organisons à la fois la solidarité interprofessionnelle entre les acteurs économiques, puis dans un second temps à renforcement et une garantie avec l'État puisque le par principe même à avec un un tels aléas quand il touche tout le monde, ça n'est plus justement aléatoire, c'est une certitude, donc ça n'est pas assurable, c'est cet objectif sur lequel aujourd'hui par cet amendement, je propose au Sénat de confirmer la volonté pour permettre, je le redis à ce qu'un dispositif puisse progressivement se mettre en place, en lien avec la profession des assureurs, monsieur le ministre, vous me l'avait glissé, j'ai vérifié également un accord est intervenu ce matin avec les compagnies d'assurance et le gouvernement sur un gel des cotisations 2021 des primes d'assurance pour un certain nombre de secteurs d'activité, dont : hôtels, cafés, restaurants je vous laisserai le soin d'ajouter les autres mais je suis allé par curiosité, voire et le ministre explique qu'il n'y aura pas d'assurance pandémie qu'il n'y aura pas d'assurance dites obligatoires, etc en fait ce qu'on appelle des captives pouvoir éventuellement être mises en place par les acteurs économiques et moi je dis qu'ils le pourront, hé bien je pense. Que cette une forme de de gifles qui est envoyé à la réflexion qui est que nous proposons et qui a été fait, le gouvernement mis en place un groupe de travail sur les risques exceptionnels, ce groupe de travail a réuni tout le monde, et j'y ai participé mais comme beaucoup d'autres, aujourd'hui il y a pas eu d'échange des conclusions. Il y a eu un état des lieux et là le ministre, alors il a le droit, mais j'appelle pas ça du dialogue, j'appelle ça une forme de mépris à l'endroit du travail collectif qui a été menée, dit il n'y aura pas d'assurance du tout, je continue de dire : c'est une erreur, c'est une faute, nous avons besoin de partager et de construire une une ligne est un dispositif qui pourrait peut-être prendre du temps mais il faut éviter de ne réserver un dispositif susceptible d'être mis en place demain casser les ce qui pourrait éventuellement faire de l'entre-soi c'est pas de l'entre-soi qu'on veut, c'est un dispositif qui puisse profiter à toutes les entreprises de France. Merci monsieur le Président, j'entends la volonté du rapporteur d'inscrire dans le PLF Les les conclusions en tous cas des dispositions que le Sénat a adopté examiner concernant la question des assurances, comme l'a dit monsieur le rapporteur à l'instant, un accord est intervenu ce matin, il prévoit un gel des des cotisations d'assurance pour le secteur de l'hôtellerie les cafés de la restauration, il prévoit aussi ces même gel pour les secteurs les plus touchés, le tourisme événementiel, la culture et le sport, je je ne fais pas la liste totale vous la, vous la connaissez à force que nous veillons à discuter des secteurs et sans et Saint-Lys, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où cela vient s'ajouter aux dispositions prises par le secteur des assurances que j'avais eu l'occasion de rappeler en première partie, la participation à hauteur de 400 millions d'euros au fonds de solidarité et je rappelle que c'est le seul secteur professionnel à l'avoir fait, le fait d'avoir mis en place un plan d'investissements dans les secteurs les plus touchés, pour un milliard 5 et enfin des des remises gracieuses commercial à leurs assurés à hauteur de 2 milliards d'euros, ce qui représente 4 milliards d'euros

un quelconque refus de la tranchée qui est celle de la prise en charge assurantiel d'une perte d'exploitation et des conditions dans lesquelles cette prise en charge pourrait être envisagée, le groupe de travail qui a été évoqué doit continuer sa réflexion, nous devons y veiller et dans l'attente, le ministre de l'Économie a annoncé tout à l'heure que dans l'attente de la refonte de ses contrats, ce qui nécessite un travail et et une analyse évidemment, nous mettrons en place un système qui permettra aux entreprises, à la fois concernés et le pouvons j'ai conscience du caractère relatif de mes propos, à cet instant, de mettre en place des provisions avec un régime fiscal particulièrement avantageux pour aider à la mise en place de provisions, c'est là l'ensemble du dispositif que nous proposons, cela m'amène à avoir un avis défavorable sur l'amendement de monsieur le rapporteur, au bénéfice de la poursuite des travaux au bénéfice aussi des avancées obtenues ce matin et qui seront complétés par le dispositif d'accompagnement fiscal des provisions pour les entreprises concernées. Monsieur Karoutchi pour une explication de vote. l'amendement du rapporteur, Monsieur le Ministre, vous dites au rapporteur, c'est une première étape, etc, poursuivant le groupe de travail et le le rapporteur général vous dit lui-même c'est bien, il y a un groupe de travail mais finalement, au bout du bout, on n'est pas associé et vous décidez le gouvernement décide sans faire un échange de conclusion avec les parlementaires, le rapporteur général ou d'autres d'ailleurs, à un moment il faut arrêter de tourner en rond, on apprend ce matin ce matin que 30 citoyens vont être tirés au sort pour définir la campagne vaccinale non mais pardon, mais c'est à un moment, il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi, enfin je veux dire, moi qui suis favorable au référendum d'initiative populaire, à un moment, je vais dire halte au feu, parce que si tout est, tout est est fait dans le tirage au sort, c'est en réalité un moyen pour le gouvernement de ne plus être responsable devant le Parlement, et c'est un moyen pour le gouvernement de se défausser de ce qui peut se passer, franchement, à un moment l'activité politique à une noblesse, c'est celle de décider de trancher et d'être responsables devant les électeurs, c'est pas du tirage au sort. je m'associe évidemment merci monsieur le président, monsieur le ministre, par rapport à vos propos, il faut savoir que les professionnels de l'hôtellerie mais et professionnelle en général réclame à ce que ce dossier de 4 textes avance mais est il n'y a pas que les professionnels de telle risques ont été touchés, il y a aussi des assureurs, les assureurs, qui veulent avoir une position claire dans l'avenir, sur comment ils interviennent quand je vois aujourd'hui que le ministre fait la promotion des des banquiers, mais il faut rappeler avec le PGE et j'en passe, les banquiers n'ont fait que gérer l'argent que vous leur avait confié depuis le départ, on vous dit qu'on sait que les assureurs savent traiter des pertes d'exploitation que des professions telles que les hôtels restaurants ne s'en remettront pas d'un deuxième confinement et un confinement qui dure, où toutes les grosses périodes vont vont être passés depuis le départ, on vous dit que c'est indéniable, on ira vers une perte d'exploitation vers ces professions-là, pourquoi vous n'avez pas confier comme vous avez confié de l'argent aux banquiers, vous n'avez pas confier de l'argent pour qu'on règle les pertes d'exploitation et de sauvegarder ces ces entreprises-là d'envoyer de l'argent dans des chômages partiels dans des sur des Ribes étranger je pense que les assureurs n'aurait pas fait ce là.

la prise de position du gouvernement il y a, je pense qu'il y a une erreur en ce moment avec ce dispositif, alors je pense qu'on va y voir plus clair dans les heures qui viennent, mais que je vais appeler peut-être intermédiaire peut-être intercalaires mais peut-être quasi définitif, le gouvernement finalement il laisse les entreprises qui peuvent faire leur affaire de d'un dispositif de prévention de précaution et finalement ils fichent la paix aux assureurs je pense que l'assurance et on l'a vu, je l'ai aussi entendu a aujourd'hui une réflexion à produire encore, elle n'est pas évidente, ça on peut entendre mais il ne faut pas que d'un côté, on a l'impression finalement que par un un jeu d'évitement, on oublie le dispositif, je vais vous dire, je pense qu'on a une responsabilité particulière, alors j'ai entendu, même la présidente de la Fédération française des assurances, expliquer que les politiques faute de décider n'avait toujours comme solution que de taxer et de faire payer des impôts supplémentaires moi j'invite la présidente. Un peu plus de retenue, je pense que nous essayons, en tous les cas de trouver des modalités par lesquelles un nouveau dispositif pourrait être trouvée construit mais ça se ça doit aussi s'accompagner de prévention de dispositif où les entreprises pourraient dans un 1er temps je dirais mieux s'organiser éventuellement constituer des réserves de précaution susceptible de c'est la question des fonds propres, voilà je mais je crois, enfin en tous les cas, sachez que notre volonté, c'est de travailler à faire des propositions, c'est pas d'éviter, c'est je pense, d'être aussi au rendez-vous, pour nous, de la responsabilité. Je vais mettre au point cet amendement, quels sont ceux qui sont en Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, l'amendement est adopté, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour la suite de l'examen des articles de la seconde partie non rattachés au crédit du projet de loi de finances pour 2021, la séance est suspendue.